La séance est reprise. La parole est à madame Annick Jacquemet pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci monsieur le président je souhaite procéder à une rectification de vote celle-ci concerne le scrutin numéro 29 sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables notre collègue Hervé Maurey souhaité s'abstenir. Merci, cher collègue acté donner de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans la vie politique du scrutin concernés nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'amendement 698 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 qui ne présentent madame Annick Jacquemet. Oui, merci Monsieur le Président, une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficient d'une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l'obligation pour l'employeur de participer au financement, en revanche, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficie d'aucun mécanisme d'aide pour pallier cette différence de traitement, l'amendement que je vous présente, au nom de Jean Michel Arnaud vient compléter l'article L 862 IV du code de la sécurité sociale, afin de fixer un 7 0 le taux de la taxe de solidarité additionnelle la TSA applicable au contrat ne bénéficiant pas d'Avantage fiscal ou de prise en charge par l'employeur de la cotisation, ce taux de TSA serait calibré de façon à offrir à cotisation identique à la complémentaire santé un Avantage équivalent à celui des salariés du privé, il y a celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable, vous l'aurez compris le présent amendement s'inscrit dans une véritable logique d'équité et de justice sociale, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président en en réalité voilà nous comprenons bien l'objet de votre demande ou ou celle de de votre collègue Jean Michel Arnaud, mais en fait, à la sécurité sociale de subir les conséquences du choix de l'employeur, parce que évidemment il y a les employeurs qui participe à ces frais et puis à ceux qui qui ne le font pas une telle réduction pourrait même je pense constituer une incitation à ne plus participer au financement de ces contrats, donc c'est un avis défavorable. Y'Monsieur le Ministre, même avis. Défavorable, donc je mais aux voix l'amendement 698 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement de la commission de 37 madame la rapporteure.

qu'à défaut d'accord avant le 1er février 2023 entre l'assurance maladie et les biologistes médicaux un arrêté fixera une baisse pérenne de cotation des actes de biologie médicale non liés à la Covid 19 devant générer une économie de 250 millions d'euros dès 2023, donc c'est en fait une contribution qui serait pérenne je, je veux dire qu'avant il y avait des protocoles d'accord entre l'assurance maladie et les laboratoires et ça depuis 2014 et ça fonctionnait très très bien seulement entre-temps on a eu la Covid 19 et les choses ont un un petit peu changé : il s'agit donc là d'une proposition qui n'a rien d'autre qu'un et un ultimatum dont l'issue est une diminution du remboursement des actes de biologie qui affecterait tous les laboratoires, et quels que soient leur taille et quelle que soit leur activité en lieu et place de cette mesure, l'amendement de la commission propose de créer une contribution exceptionnelle assis sur les sommes versées en 2021 par l'assurance maladie et je voudrais rappeler qu'en 2021 hé bien ce remboursement s'élevait à 2 7 milliards d'euros et donc ce serait versée par l'assurance maladie, enfin cette somme versée à la de l'assurance maladie au laboratoire seraient prises en compte à charge du dépistage de la Covid 19 cette contribution serait seulement du en 2023 en contrepartie du chiffre d'affaires réalisé par le secteur en raison de la crise sanitaire, elle serait plus juste car acquitté en proportion des sommes reçues de l'assurance maladie et en 2021, le remboursement donc devrait s'élever avec un moment un amendement qui propose de fixer le taux de la contribution à 9 17 % hé bien ça généré un produit de 250 millions d'euros. d'euros. Un rapporteur, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la rapporteure générale votre amendement propose de de créer une contribution exceptionnelle de laboratoires de biologie médicale avant toute chose, il faut rappeler que l'investissement des biologistes médicaux durant la crise sanitaire a été totale, que, en conséquence de cet engagement, leur chiffre d'affaires a lui aussi augmenté en passant de 5,1 milliards d'euros à 9 4 milliards d'euros entre 2000 19 et 2021 et que, au même moment, le taux de rentabilité des des biologistes médicaux et a lui aussi augmenté, il est passé à plus de 30 % contre 16 % en 2019 la solution proposée par le gouvernement n'est pas sorti tout à fait du chapeau puisqu'elle a été négocié avec la CNAM et les syndicats de de biologie, ces discussions ont d'ores ont d'ores et déjà démarré, c'est la raison pour laquelle la solution qui est proposée par le gouvernement, nous y restons favorables et que nous avons un avis défavorable sur la solution exceptionnelle que vous proposez pour privilégier une solution plus durable. Merci, parce que je sors.

il y a une imposition sur un surplus de gains, mais effectivement, on peut espérer que le Covid ben va ne va pas générer autant de dépense et je pense que la solution de madame, le rapporteur général est beaucoup plus juste et en tout cas cette solution de gouvernement, elle pourrait gêner des petits laboratoires puisque c'est quelque chose qui se perd, se perpétuer dans l'avenir et et donc elle pourrait gêner les petits laboratoires, notamment ruraux, merci, merci madame Jacques, mais. Oui, monsieur le président, moi aussi je soutiendrai cet amendement pour les mêmes raisons, j'ai été aussi contacté par des laboratoires qui sont situés en milieu rural parce que je suis élue dans un département où il y a beaucoup de petites communes et puis où la ruralité, très présente et ils sont très inquiets de ce qui est prévu par le gouvernement, ils ont de gros investissements à faire aussi pour rester au niveau, et pour rester compétitif avec les gros groupes de laboratoire, donc je soutiendrai aussi cet amendement, je vous remercie. Monsieur le Président, nous allons évidemment soutenir l'amendement présenté par par la rapporteure, mais je voudrais ajouter, Monsieur le Ministre, que si vous vous vouliez à tout prix récupérer de l'argent pour faire en sorte que le PLFSS 2023 sont moins dramatique que celui de 1022, il aurait peut-être fallu à l'époque où vous avez mis en place les tests et les vaccins, penser à faire participer d'autres organismes qui la sécurité que la sécurité sociale et en particulier les organismes qu'on appelle au calme, s'ils n'ont pas participé du tout puisque le gouvernement a décidé, c'était pris en charge intégralement, c'est regrettable mais c'est plutôt de la faute du gouvernement que de notre faute à nous et du que de la faute des laboratoires femme biologique en particulier. Merci, cher collègue, Madame Guigou Oui, moi je vais également soutenir la l'amendement de la présidente de la fin de la rapporteure et de la commission des affaires sociales, je pense qu'il est quand même plus juste de prélever une taxe sur quelque chose d'exceptionnel que d'instaurer une baisse des tarifs pérenne en sachant que, voilà le la période Covid est derrière nous, enfin en tout cas on le. monsieur le président, Monsieur le Ministre, oui les, les, les chiffres sont clairs, vous les avez exposé, Monsieur le Ministre, le chiffre d'affaires a presque doublé la marge aussi et donc c'est une argumentation suffisamment clair pour voter l'amendement de la rapporteure générale, je vous remercie. Merci, cher collègue, donc oui, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, simplement pour rappeler que les les les chiffre que je vous ai présenté ne nous semble pas être la simple résultante de l'épisode de Covid mais qu'il y a bien une tendance, notamment à la concentration dans le marché des biologistes médicaux qui va conduire assez naturellement à à une progression de la marge qui appelle donc des, des, des efforts complémentaires mais ces efforts complémentaires ne sont pas imposés, ils sont négociés et comme j'ai dit tout à l'heure, les discussions entre la CNAM les gestes médicaux ont démarré. Merci, monsieur le Ministre, donc je mais on voit cet amendement 37 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté nous pas sur l'article 9 le 38 de la commission madame la rapporteure. Un amendement rédactionnel. Monsieur le Ministre, favorable, favorable, il y a pas d'opposition ni abstention c'est adopté, nous poursuivons avec 272 Monsieur Chassaing. monsieur le Président, donc cet article, si vous voulez ce cet amendement, c'est pour les médecins retraités qui ne font pas beaucoup de remplacement, mais ils ne souhaitent pas payer la retraite car en effet ce paiement est à fonds perdus, on en a parlé,

défini à l'article L 642 cas de du groupe, code de la sécurité sociale, pour un coût moins important, mais il y a des cotisations quand même, mais pour cela, leur chiffre d'affaires doit être très inférieur à trois très ce qui réalise très peu de remplacement donc ce seuil est défini par décret, il serait nécessaire pour combler une partie de la pénurie des médecins de porter ce plafond à 40000 euros ce chiffre d'affaires bien sûr sans condition à la Caisse autonome de retraite des médecins français qu'on viendrait-il donc de modifier le seuil des rémunérations issu de l'activité de remplacement, c'est ce que demande cet amendement. Oleg madame la rapporteure. Oui, actuellement, le plafond de revenu est fixé à 19000 euros, alors s'il peut être envisagé comme vous le proposer de relever ce seuil, le dispositif comparables au régime des micro-entreprises et réservé aux médecins remplaçants et aux étudiants en médecine qui assure des remplacements à titre occasionnel. Ce qui dégage par conséquent des revenus assez faibles, et pour lesquels le bénéfice d'un allégement des démarches déclaratives et le plus important concernant les médecins en cumul emploi-retraite, il me paraîtrait plus pertinent, je pense qu'on a eu d'ailleurs le débat de leur permettent de s'ouvrir des droits en contrepartie des cotisations de retraite versée à défaut de pouvoir le prévoir, par le biais d'un amendement parlementaire, j'estime suffisant le dispositif que nous avons pris tout à l'heure de l'article 7 sexy qui exonère de toute cotisation vieillesse due au titre de 2023, les médecins en cumul emploi-retraite justifiant de revenus inférieurs à un certain niveau, nous devrons avoir dans les mois à venir, un débat sur ce sujet important au regard des enjeux de lutte contre la désertification médicale et de soutien à l'emploi des seniors dans cette attente, j'émets un avis défavorable à cet amendement. Merci monsieur Ministre même ma vie. Défavorable dont je mets au voile de sauf il est retiré l'amendement est retiré, le trente-neuf de la commission Madame Lamy le rapporteur. Oui, bien que pertinente sur le fond les disposaient les dispositions relatives au régime de responsabilité des médecins régulateurs du service d'accès aux soins n'aurait d'effet ni sur les recettes, ni sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et notre et n'entrent donc pas dans le Champ des lois de financement de la Sécurité sociale, telle que définie par la loi organique, cet amendement vise donc à supprimer cette disposition dans l'attente d'un véhicule législatif plus adapté. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, s'agissant de de l'extension de, de, d'un dispositif à à une population plus large, il a semblé au gouvernement que que cette disposition pouvait avoir un impact en recettes ou en dépenses, c'est la raison pour Alcatel, elle est inscrite dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, de retirer cet amendement et de laisser le constitue le Conseil constitutionnel jugé le moment venu si oui ou non elle est conforme à la Constitution. Merci, c'est un retrait sinon défavorable. Il est maintenu, donc je le mais aux voix l'amendement trente-neuf de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté je mais on voit l'article 9 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté à à l'article 9 bis de prise de parole Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, quelques mots pour vous dire que nous nous abstiendrons sur cet article 9 bis désormais situées dans la partie recettes, en effet, nous avions à neuf excusez-moi.

quelques mots, je recommence pour pour vous dire que nous nous abstiendrons sur cet article ne vise désormais situées dans la partie recettes, en effet, nous avions proposé un amendement qui a été déclarée irrecevable pour abaisser le seuil de déclenchement de la clause de de sauvegarde à 23 6 milliards d'euros pour le montant plafond, dit M, à savoir pourtant sur les médicaments, au lieu des 24 6 milliards inscrits initialement, j'ai bien encore en tête les propos notamment du président l'an dernier, expliquant que le déclenchement de la clause de sauvegarde n'était pas par nature pas censée intervenir mais le contexte sanitaire actuel conjointement, celui de la croissance du médicament va sans doute au contraire dynamiser le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques en le situant désormais dans la partie recettes, ce qui nous paraît pertinent, nous proposions d'offrir un peu plus de marge financière, à notre système de protection sociale en mettant un peu plus à contribution les entreprises pharmaceutiques, qui je le rappelle, se porte vraiment très bien, pour ne citer qu'un exemple, directeur de Sanofi Paul Hudson perçoit un salaire d'environ 12 millions d'euros annuels faisant de lui l'un des patrons les mieux payés du CAC 40 le bénéfice Net de ce grand laboratoire a connu une hausse de 340 pour 100 en 2020, passant à 12,3 milliards d'euros les dividendes ont connu leur 28ème année consécutive de hausse, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros, et ce malgré l'échec sur le vaccin contre contre la Covid 19 parallèlement à ces produits profits colossaux, Sanofi a poursuivi sa politique de licenciement aussi ne nous sommes pas exagérer de demander un effort sur la contribution de ces entreprises en cas d'évolution de leur chiffre d'affaires, c'est pourquoi nous voulions réévalué à la baisse et non à la hausse, comme proposé par cet article. Ou par l'amendement qui va suivre, de notre collègue Folio le montant, M. je vous remercie. Merci si cher collègue Monsieur Mignon. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, à l'occasion du Conseil stratégique des industries de santé de 2021, le président de la République avait annoncé plusieurs mesures visant à faire de la France, la première nation européenne innovante et souveraine en santé, c'est sur ces mots, le plan Innovation Santé 2030, prévoyez plusieurs actions visant à renforcer nos capacités de recherche biomédicale à investir dans les biothérapies et dans la bioproduction de thérapies innovantes de faire de la France, selon encore ces mots le pays leader en Europe sur les essais cliniques ou encore de soutenir l'industrialisation des produits de santé lors du sommet choose, France 2022, le président a rappelé le caractère stratégique de l'industrie pharmaceutique ce PLFSS 2023 contient des mesures qui contredisent complètement les discours du président de la République en accroissant considérablement la pression économique sur l'industrie pharmaceutique, 2 principaux éléments illustrent cette réalité j'irais pas au delà, mais dans le cas des débats, on pourra continuer un montant d'économies demandées au secteur du médicament à plus de 800 millions d'euros sous forme de baisses de prix qui s'ajoute au montant déjà imposé depuis de nombreuses années et puis une charge pesant sur les entreprises pharmaceutiques du fait de la clause de sauvegarde dont le rendement prévisionnel pour 2023 et c'était, il est 2 milliards 400 millions d'euros, plus 800 millions 3 milliards de plus tout le reste qui existe depuis plusieurs années, ces éléments portent atteinte, monsieur le Ministre à la pas citer d'innovation des entreprises et en selon moi et selon nous, nous au niveau d'autres groupes, un signal négatif aux entreprises innovantes. Merci, cher collègue, le l'amendement 311 Madame Micouleau. Merci monsieur le président, la clause de sauvegarde des médicaments et de une contribution qui a pour objectif de maîtriser les dépenses courantes de ces produits dans le cadre de des lois de financement de la Sécurité sociale, il est proposé de conserver dans cet amendement, dans l'attente de du rapport de la mission de financement, la régulation des produits de santé, les modalités actuelles avec le calcul de la clause de sauvegarde. Merci monsieur le président, monsieur le Ministre, chers collègues, je comprends évidemment l'intention de derrière cet amendement est en effet important de veiller à ce que l'inclusion des médicaments qui seraient acquis par Santé publique France soit bien prise en compte dans la définition du montant, M. pour quelle note monte pas artificiellement le montant de cette contribution toutefois puisque la clause de sauvegarde a vocation à permettent de réguler les dépenses d'assurance maladie relative à l'ensemble des médicaments et puisque le gouvernement a reporté cette évolue sur la pelouse de 1024 qui sera appelé en 2025 la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

peut ajouté dans la balance, les 7 milliards et demi d'euros qui seront consacrés par France 2030, au développement de notre industrie souveraine en santé, ce n'est pas tout à fait l'objet de cet amendement, mais c'est néanmoins un élément que je voulais apporter dans dans la discussion, s'agissant de la clause de sauvegarde

que nous traversons, après discussion avec le secteur, il a été décidé de faire évoluer la la la structure, la la la la la composition de la clause de sauvegarde qui ne sera plus plus exclusivement fondée sur le prorata des chiffres d'affaire mais inclura à hauteur de 30 % la prise en compte de l'évolution du chiffre d'affaires des des entreprises, nous allons examiner enfin vous allez examiner une série d'amendements qui visent à à réduire la la clause de sauvegarde ou en en minimiser l'impact, le gouvernement sera défavorable à l'ensemble de ces amendements mais j'essaierai néanmoins d'y répondre point par point, quant à l'amendement en question, je veux pas reprendre les excellents arguments de Madame la rapporteure et et c'est donc un avis défavorable. Merci donc je la mais on voit le 311 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 4 amendements en discussion commune le 721 madame Oui, là aussi, Monsieur le Président, cet amendement Paul sur la clause de sauvegarde et la place des Medhi médicaments génériques par définition la clause de sauvegarde est en fait pour réguler pour réguler le marché du du du médicament, les génériques sont déjà des produits qui ont été largement réguler à Bakou par rapport aux molécules existence et, en conséquence, c'est la régulation sur la régulation, c'est la raison pour laquelle même semblé peut être intéressant d'exclure

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oui. La crise de pandémie que nous en montrer combien il était essentiel d'avoir une forme de sécurité pour ne pas dire de souveraineté au regard de, de, de, des médicaments et nous avons vu toutes nos faiblesses en la matière, force est de constater qu'en 30 ans, l'industrie française du médicament est passé du du 2ème rang européen au 5ème rang européen, c'est-à-dire un véritable déclassement et ceci est la conséquence, finalement, de la stratégie qui a été celle au fur à mesure du vote des différents projets de loi de financement de la Sécurité sociale, de se servir de l'industrie de médicaments comme une variable d'ajustement à certains égards pressuriser les prix et, du reste, ne faisant aucune différence entre les médicaments fabriqués en France, dans le cadre d'un schéma d'une certaine souveraineté et ceux qui qui était venant de l'étranger aujourd'hui nous sommes dans cette situation et et nous continuons et et du reste ce que l'on peut constater, comme l'a fort justement souligné notre collègue tout à l'heure et et certains autres orateurs, nous sommes dans une situation qui est une situation qui devient très difficile pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique alors que le projet de loi de le financement de la Sécurité sociale pour 2023 fixe une croissance de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie à 3 scènes % et que le montant de, de, de 2022 États, fixé à 24 véhicules

dans ce cadre, il nous appartient de veiller à c'est c'est le sens de cet amendement à faire de telle sorte que en ce qui concerne les dépenses de produits de santé, donc 1,7 % sur les médicaments soient prises en compte à à la à la hauteur de ce qu'il représente sur un plan économique et en termes de souveraineté. Merci, cher collègue Madame la rapporteure sur ces deux amendements. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, concernant l'amendement 528 de Monsieur Savary en exonérant de la clause de sauvegarde les médicaments génériques biosimilaire hybride et mature, cet amendement permet de protéger les spécialités génératrice d'économies, il contribue à rééquilibrer la clause de sauvegarde afin de mieux faire porter l'effort par les médicaments, responsable de la forte croissance des dépenses de produits de de santé comme elle l'avait fait l'année dernière, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve d'une rectification consistant à tenir compte en effet de cette exclusion sur le montant, pour ne pas affaiblir artificiellement la clause de sauvegarde la rectification a bien été réalisé, donc c'est un avis favorable sur l'amendement mille sept de monsieur Folliot alors à l'inverse, en augmentant le le montant, M. cet amendement diminue évidemment la clause de sauvegarde éventuellement dues par les entreprises au titre de 2023 plusieurs modifications ont déjà été apportées au texte à l'Assemblée nationale pour tenir compte de l'inquiétude des industriels, notamment par l'ajout d'un d'un plafond de plus, la clause de sauvegarde devient progressivement l'un des principaux outils de régulation des dépenses de produits de santé, et ce depuis longtemps, je partage les propos de nos collègues à la mi-longs et de notre collègue Folio, sa répartition a été revu pour mieux cibler les les médicaments en forte croissance, donc sur l'amendement mille sept c'est un avis défavorable. Monsieur le Président, peut-être quelques éléments d'abord en réponse à monsieur le sénateur, Folio pour dire que dans les négociations de de de prix qui sont conduites sur les médicaments, il y a évidemment de la latitude pour faire une une différence entre les les médicaments qui sont produits en France dans le dans nos territoires et les médicaments qui sont produits à l'étranger, mais je veux simplement une nouvelle fois rappelé que le prix n'est pas la seule dimension de notre politique industrielle et et je citais tout à l'heure, les 7 milliards et demi qui sont inscrits dans France 2030 ils sont gérés par l'des pays et qui vont contribuer à à nous aider à bâtir cette cette souveraineté dans la régulation, il y a aussi la question des volumes qui sont adressées dans la partie IV du du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec les rendez-vous de prévention à un certain nombre d'âge de de la vie qui vont permettre de de maîtriser une partie des volumes et de et de la dépense et puis enfin quand tu les prix, l'action sur les prix et l'action sur les volumes n'a pas suffi, il reste comme l'a dit le rapporteur, la clause de sauvegarde qui est le dernier mécanisme de de régulation de nos dépenses en santé et c'est la raison pour laquelle nous considérons avoir trouvé le bon équilibre et que les les 2 propositions qui qui ont été présentés, même si on comprend bien l'intention, celle d'exclure les génériques qui font l'objet de discussions sur les prix qui sont relativement serrés et celle d'un d'un relèvement du du montant, M. qui déclenche la clause de sauvegarde, on comprend bien d'où ça vient mais ça fragiliserait cet édifice, ceci étant dit, cet édifice n'est pas idéal, puisqu'on a besoin de cette clause de sauvegarde qui est activé depuis 2 3 ans pour faire la régulation et que ça n'est pas satisfaisant de d'avoir une mesure d'or générales pour réguler la dépense en santé et c'est la raison pour laquelle nous avons avec un un amendement de de la rapporteure générale à l'Assemblée un article Dister au texte qui vous est soumis : Ce soir, qui permettra d'ouvrir largement la discussion sur la régulation des dépenses en santé et plutôt, je dirais que d'ajuster ou de fragiliser la la clause de sauvegarde d'embrasser très largement tous ces sujets, donc un a un avis défavorable sur ces 2 amendements. Et Monsieur Savary. Oui, Monsieur le Ministre, dans le cas du Plfss est devenu complètement opaque où on on met des tout et Alain Milon avait raison : des taux de progression, par exemple, pour cette année par rapport à la même époque l'an dernier entre deux dans la réalité des choses le taux, elle a été déjà largement dépassé de cette année 2022, et en conséquence, arrivé par exemple à peu près au mois de novembre, les médicaments qui vont être vendus vont automatiquement. Allez dans la clause de sauvegarde de quand il y a un choix à faire, comme ce sont des entreprises européennes, ben ils vendent plus à la France, faut pas s'étonner après qu'on ait des problèmes de médicaments, donc c'est antinomique par rapport à la souveraineté, c'est la raison pour laquelle il faut peut être voir le dispositif alors quand est-ce qu'il nous a expliqué dans le PLFSS franchement il y a plus rien y comprendre, mais la clause de sauvegarde, c'est devenu une taxation a, il y a, il y a dérive la plus complète et puis il faut agir, surtout sur les prescriptions hors les efforts sur les prescriptions sont pas d'une redoutable évidence et c'est là qu'il faudrait faire, parce que là vous pénalisez vous pénaliser les, les, les entreprises pharmaceutiques, ce que je comprends bien, mais elles, elles vendent les médicaments qui ont été prescrits. prescrits. C'est pas elle qui vont boîtes de paracétamol, si il a une préinscription que d'une boîte, donc il est peut-être celui qui prescrit qu'il faut voir et là où là on sait, on l'a déjà largement débattu notamment avec Jean Marie il y a la pertinence des actes les prescriptions pour lequel il y a des efforts véritablement à faire en attendant merci madame le rapporteur, de donner un avis positif, sur mon amendement, puisque les génériques, les bio-séminaire les les médicaments matures, ils ont déjà été largement taxé, hein, si on veut qu'on continue à trouver des mendier des médicaments matures sur le marché, il faut peut-être arrêter un peu de les taxer quand même quoi, c'est la raison pour laquelle j'avais proposé ça, donc je retirerai pas mon amendement, il faut, il faut faire une discussion mais attention, les labos collègues n'ont pas le même discours que celui que vous nous tenez. Merci, cher collègue, mais les lustres. Oui, simplement monsieur le le le sénateur là la politique du du prix du médicament, elle n'est pas là uniquement pour équilibrer des des comptes dans la discussion chaque année sur le projet de loi de financement de la la sécurité sociale, elle est là aussi, elle a été conçue, elle a été, elle a été conçue initialement pour que le médicament soit accessible pour nos concitoyens, évidemment que, il y a des discussions qui ont lieu et vous avez raison sur les génériques, c'est particulièrement serré et parfois dans nos dans dans les les territoires dans lesquels l'industrie pharmaceutique à une implantation assez forte, ça peut poser des questions sur cette politique du prix et et ses limites, notre politique de de de souveraineté, elle ne s'arrête pas à la clause de sauvegarde, puisque je rappelle pas le chiffre de de France 2000 30 mai on peut rappeler également les la baisse des impôts du de de production qui vont permettre là aussi de conforter les industriels français

Monsieur le Ministre, vous savez que dans l'industrie du médicament il y a un élément qui est un élément essentiel, c'est la recherche et que c'est long, c'est difficile, c'est compliqué et ça nécessite des moyens et que si on veut avoir une industrie pharmaceutique performante, il faut-il qu'elle puisse avoir un minimum de marge sur les médicaments que l'on vend aujourd'hui pour pouvoir investir dans la recherche s'étonne un jeu est un élément essentiel, et je trouve dommage que dans vos propos, vous ne mettiez pas en avant ces éléments-là parce qu'il faut essayer d'avoir une stratégie globale et et, in fine, et que tout ceci a pour conséquence ce déclassement auquel je faisais référence au tout à l'heure et le fait que nous perdions des places dans l'industrie européenne et nous retrouver maintenant au 5ème rang bientôt 6ème ou 7ème et ça c'est quelque chose de catastrophique au de l'un des, des éléments de souveraineté, parce que je ne parle même plus aussi de questions de souveraineté nationale parce que c'est les mêmes questions qui se posent à l'échelle européenne, mais quand on sait tout le temps qu'il faut pour développer un médicament, hé bien je crois qu'il faut avoir une vision globale et que cette vision globale passe par la prise en compte des éléments industriels après par rapport à des propos, qui j'ai j'ai entendu tout à l'heure de certains collègues au regard des actionnaires, et cetera, de l'industrie du médicament c'est pas partout pareil, il existe de certains nombres de groupes de groupes pharmaceutiques qui sont détenues par des fondations et pour lesquels l'argent qui peut être gagné dans ce cadre-là et investi dans le but social de cette fondation, et ça c'est quelque chose, et qui est une réalité, une réalité de terrain et quand en plus, ces groupes investissent dans les territoires depuis des décennies pour essayer de développer tout un microcosme de toute vertueux de développement économique et territorial, hé ben c'est dommage que par le biais de décisions comme ça trop rapide et trop arbitraire hommes mettent en péril toute une industrie et et et à certains égards, développement et les perspectives d'un territoire.

l'emprise des laboratoires sur à la fois le prix des médicaments et la la politique du médicament avec des pénuries qui sont entretenus, c'est comme si il y avait rien, moi je ne sais pas, mais alors que les pénuries de médicaments se multiplient dans notre pays et il y a eu des rapports qui sont extrêmement intéressant du Sénat transpartisan qui ont démontré ces ces pénuries entretenues que même le paracétamol est un produit en rupture, je crois qu'au contraire on a, on a vraiment besoin d'en tirer les enseignements est-ce que les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que le gouvernement se prive d'un outil important c'est d'avoir une maîtrise publique et une souveraineté hé oui mes chers collègues, c'est pas ça existe dans des tas de pays qui ne sont pas des pays communistes, ça se passe au Brésil, ça se passe, il y a des expériences en Inde il y a des expériences en Afrique, en Suisse, et même aux États-Unis, mais au au moins ils ont un outil ou quand il a besoin d'un médicament, quand il a besoin d'un vaccin, hé bien ils peuvent effectivement intervenir, ça se passe d'ailleurs dans notre pays avec la le qui dispose d'une pharmacie centrale qui peut produire des médicaments au seul enfin des des des hôpitaux de la PHP et on pourrait généraliser mais vous vous refusez tout ça et on est en train de nous faire finalement le le les les qualités extraordinaires des laboratoires pharmaceutiques qui ne se font absolument pas des milliards d'euros d'euros de bénéfices et surtout qui ont engrangé des dividendes au détriment parce que la recherche, mon cher collègue, elle est, elle est faite et mais elle est faite par des fonds publics et après les brevets sont détournés par le privé, alors un peu d'essence. Monsieur le Président, je pense que je vais encore, je crois qu'il y est un peu plus notre collègue Laurence Cohen, je voudrais quand même quand même lui rappeler qu'hier dans mon intervention, j'ai quand même dit Monsieur le Ministre, c'est important que lorsqu'un laboratoire avait l'autorisation pour son médicament par la Haute autorité de santé, il lui fallait ensuite négocié son prix avec le CE, PS et que généralement, les délais sont de 18 mois avant qu'ils obtiennent, après l'autorisation le le la la mise sur le marché, or 18 mois c'est le contraire de ce qui se passe en Allemagne, où ces trois mois en Angleterre où c'est de moi et caetera, on a des délais tellement long que finalement les médicaments sont plus facilement vendu en Allemagne ou en Angleterre, parce que les délais sont nettement plus court, ça c'est le 1er point, je voulais dire à notre collègue Laurence et puis quand on discute avec les laboratoires pharmaceutiques, quel qu'il soit avec le OM en particulier puisque c'est un ça risque de choquer un peu plus Laurence mais enfin quand on discute avec les les grands laboratoires pharmaceutiques, ils ne le disent tous la même chose, on est pas contre le fait de participer à la solidarité nationale, bien au contraire, on souhaite le faire, on souhaite le faire au maximum de nos possibilités, à une condition,

OK, ils ont fait des chiffres d'affaires plus important, mais c'est le pôle l'année prochaine on leur demandera peut être 4 milliards ou 2 milliards le fait ce qu'ils demandent, eux, c'est d'avoir une visibilité, ne serait-ce qu'une visibilité sur les 5 ans du mandat présidentiel, d'où la loi que j'ai réclamé hier une loi de programmation sur la santé, sur les 5 ans du mandat présidentiel de manière à ce que chacun sache où il va et en particulier la avoir enfin qui sont prêts à participer à la solidarité nationale. Mes chers collègues, je mais aux voix l'amendement 528 avec un avis favorable de la commission d'avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le président, c'est cet amendement vient mettre en cohérence de façon pérenne les modalités de calcul du plafond de versement de la contribution avec le périmètre de cette taxe sur la base du chiffre d'affaires des produits remboursables nets des différences des différentes remises visé par l'article L-1138 10 du code de la sécurité sociale, je voudrais quand même rappeler que cette pérennisation de cette mise en cohérence était nécessaire pour la protection des petites entreprises innovantes en France merci. Merci l'amendement 16 Madame Bonfanti Dossat. Afin d'assurer la souveraineté en matière du médicament ce que prône le gouvernement et de sécuriser l'approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une 3ème tranche en suce de la progression du chiffre d'affaires. Merci, cher collègue, le 331 madame Lassaad. Il est proposé que la contribution due par chaque entreprise redevable au paiement de la clause de sauvegarde soit déterminé à concurrence de 50 % au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L 138 11 et à concurrence de 50 pour 100 en fonction de la progression de son chiffre d'affaires cette évolution permettrait de remédier au déséquilibre de la régulation macro-économique au détriment des produits les plus matures et des génériques dans la mesure où certaines classes de médicaments pèse plus fortement que les autres dans la dynamique des dépenses d'assurance maladie et elle permettrait également de tirer les leçons de la crise Covid 19 en préservant la capacité d'approvisionnement du marché français, notamment pour les médicaments anciens. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur l'amendement 312 de Madame Micouleau en pérennisant le plafond exceptionnelles mises en place pour 2023 afin de répondre à l'inquiétude des industriels cet amendement risque d'affaiblir durablement le le dispositif, le code de la Sécurité sociale prévoit déjà un plafond, certes moins favorable à 10 % du chiffre d'affaires total relatifs aux médicaments mais j'espère que dans les années à venir, le dispositif sera repensé et qu'on pourra donner un peu plus de visibilité aux entreprises mais j'y reviendrai sur sur l'article 9 terre sur les amendements 16 et 331 la réforme de la répartition, la clause de sauvegarde porter par cet article permet déjà de mieux faire porter l'effort par les spécialités en forte croissance Responsable du dynamisme des dépenses, elle a été modifiée pour tenir compte des inquiétudes, des industriels, il ne paraît pas souhaitable y revenir maintenant de plus le droit de l'Union européenne ne permet pas de taxer davantage les entreprises produisant ailleurs qu'en France, donc c'est un avis également défavorable de la commission sur ces deux amendements. Le 331. Aussi,

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix l'amendement 331 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 470. Madame madame

de la clause de sauvegarde M. avec l'assiette de la clause de sauvegarde, soit le chiffre d'affaires des produits remboursables nets des différentes remises mentionnés à l'article L 138 10 du code de la sécurité sociale, afin d'assurer la proportionnalité de cette pénalité. Merci madame la rapporteure. la commission souhaite que ces majorations soit bien proportionnelle à l'importance de chaque entreprise dans les dépenses d'assurance maladie, elle a donc jugé souhaitable de tenir compte des remises verser dans leurs calculs et a émis sur cette sur cet amendement, un avis favorable. Favorable. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, cette proposition qui consiste à indexer sur un chiffre d'affaires Net des remises revient à minorer la majoration proposée cette majoration est proposé dans le projet de loi que vous examinez à à 0,0 0 5 % du chiffre d'affaires et elle est en août plafonner de manière à ce qu'elle soit en effet proportionnée et je vous rappelle l'enjeu de cette majoration qui est de nous assurer que les entreprises respectent les délais de déclaration et correction de qui sont par ailleurs allongé par la présente mesure de façon à ce que la procédure soit fluide et donc à garantir de la visibilité aux entreprises qui doivent provisionner dans leurs comptes, c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Merci donc je le mais voit le 470 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté 4 amendements en discussion commune dont 2 identique tout d'abord le 284 monsieur Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement qui vise à créer une clause de régulation des dispositifs médicaux en lieu et place du régime de la clause de sauvegarde, penser à l'origine pour le secteur du médicament loin de vider évidemment le mécanisme initial sa substance, il s'agit essentiellement d'une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l'ambition de la France en matière d'innovation à l'occasion du CSIS, 2021, le président de la République a exprimé son souhait qu'un signal fort soit adressé au secteur des dispositifs médical, le secteur a fortement contribué à l'effort de lutte contre l'épidémie de la Covid 19 et cette crise a révélé l'importance d'avoir un tissu industriel médical fort sur notre territoire, actuellement les dispositifs médicaux se voient appliquer une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur les le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traitée avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux appliqués aux médicaments même modèle économique même processus technologiques etc et donc proposé de créer un régime distinctes en ajoutant un mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux aides adaptées au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, ETI et qui, et qui sanctuarise les dispositifs les plus innovants qui représente à peine 1 % en valeur des montants remboursés cette exception temporaire, permettrait de préserver des nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter dans un 1er temps une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché afin de répondre aux besoins d'une population cible, qui ne bénéficiait pas auparavant d'une telle innovation et j'en profite pour dire que le 282 à la suite du 284 et défendu. D'accord, merci beaucoup,

Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement vise à introduire une progressivité dans la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, c'est-à-dire le montant, M. ce à quoi je suis favorable également exemptés évidemment entièrement les dispositifs innovants pendant 3 ans, je comprends bien sûr le souhaite protéger

Oui, monsieur le président, c'est absolument le même amendement et je suis flatté d'avoir présenté un amendement identique à celui de Madame, la rapporteure je sais au moins que pour celui-là, elle me donnera un avis favorable. C'est vraisemblable, madame la rapporteure sur les 284 et 282. qui ne sont pas souvent responsable des croissance des dépenses et qui sont indispensables néanmoins aux patients en conséquence, la commission a émis un avis défavorable, par contre, un avis favorable sur les amendements 283 et quarante la commission souhaite en effet introduire une progressivité de la fiscalité des dispositifs médicaux en cas de dépassement du montant Z, sur le modèle de la clause de sauvegarde du médicament. merci Monsieur le le président s'agissant de la clause de sauvegarde Z pour les dispositifs médicaux et non plus pour le pour les médicaments simplement rappeler que cette clause de sauvegarde n'a pour le moment jamais été activé et que il n'y a donc pas lieu pour les industriels qui ont été évoqués dans les débats de s'en inquiéter, à ce stade qu'elle est plafonnée à 10 % du montant des robots, des remboursements et puis enfin, et c'est peut-être le meilleur argument puisqu'il vient du sénateur Milon lui-même, s'agissant d'une clause de sauvegarde qui a été inscrite ou ou adopté dans le cadre du de la loi de financement de la Sécurité sociale 2020 pour donner suffisamment de lisibilité aux acteurs, peut être qu'on vient-t-il de la maintenir en l'état, et c'est la raison pour laquelle la position du gouvernement sur ces amendements, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défaveur. Merci, monsieur le Ministre, donc je mets aux voix le 284 avec 2 avis défavorable qui est pour. Il est retiré de 282 aussi retiré, donc je mets aux voix les amendements 40 et 283 celui de la commission et de de 183 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés le 744 monsieur le ministre. Rédactionnel madame la

Merci Monsieur le Président, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments a été mis en place pour compenser les dépenses engendrées par la promotion des médicaments remboursables par les industriels, pourtant en assurant la promotion des biosimilaire, les laboratoires pharmaceutiques contribue non seulement au bon usage de ces produits, mais ils les encouragent avec le recours à la place des médicaments de référence et génère ainsi des économies pour le système de santé, les biosimilaire ayant un prix, environ de 30 % inférieur au prix des médicaments de référence, la mise en place d'un mécanisme d'abattement de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments permettait permettrait, pardon, de reconnaître la contribution de l'activité de promotion des bio-similaires aux économies, comme cela a déjà pu être fait dans le cadre de la promotion des médicaments génériques, ainsi, cet amendement vise à instaurer une extension de l'avancement de vagues, taxe sur la promotion des génériques au biosimilaire. Merci le 450 Monsieur Chassaing. Défendu merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ces amendements Vista à créer un abattement à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments pour les bio-similaires si l'intention de de cet amendement et de soutenir le déploiement des biosimilaire et si c'est souhaitable, il est préférable de ne pas ajouter une nouvelle niche fiscale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a ouvert le cadre de la délivrance des bio-similaires, ce qui semble une voie à privilégier, il convient d'approfondir les possibilités de substitution en faveur des biosimilaire ce qui sera une source d'économie importante pour l'assurance maladie, néanmoins, pour ces raisons, c'était une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable pour ces amendements.

Monsieur le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à réduire le taux de contribution des ventes en gros à 1 % afin de dégager les moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de compenser en partie les difficultés du secteur qui, une mesure d'essentiel pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France, et seul vecteur pour livrer quotidiennement tous les médicaments dans les conditions optimales au 21000 pharmacies sur l'ensemble du territoire, la profession n'a pas de marge de valeur d'action pour pallier à cette situation, elle évalue les conséquences économiques de l'inflation et les pertes de l'exploitation des années 2021 et 2022 à 60 milliards d'euros, il s'agit d'une profession répartis bon sur l'ensemble du territoire 12000 personnes et donc consciente de l'effort national en faveur de la sobriété énergétique, le secteur envisage bien sûr d'investir dans ce domaine, c'est pourquoi la baisse de la contribution sur les ventes en gros ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demande au volley indispensable cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s'applique aux chiffre d'affaires et donc pour sa structuration par son taux, elle est devenue totalement obsolète,

Ces 267 donc on peut considérer qu'il est déjà défendu. Le 527 identique Monsieur Savary défendu merci le 1017,

la répartition a déjà bénéficié de mesures de soutien à l'an dernier une amélioration de de leur marges une réduction du taux de la contribution passer l'an dernier de 1 75 % hein et demi et une rémunération additionnelle sur les produits de la chaîne du froid par le biais d'un forfait à la boîte, mais à présent c'est l'inflation qui les place dans une position financière difficile puisqu'elle leur a creusé un gouffre financier de 43 millions d'euros dans le secteur d'ici à la fin de l'année, du seul fait que les grossistes répartiteurs ne peuvent répercuter la hausse des prix sur les prix des médicaments remboursables, la taxe étant assise sur le chiffre d'affaires ne tient pas compte de ces fluctuations de la rentabilité en diminuer en diminuer le taux serait un ballon d'oxygène pour le secteur, c'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur les amendements

néanmoins personnel et afin de soutenir le secteur je crois qu'il serait possible d'aller jusqu'à 1 % sont des c'entreprise qui assure une mission de service public et on est bien content de les trouver pour apporter livrer chaque jour les médicaments dans toutes les pharmacies de France et de Navarre, J'ai perdu mon mon pommeau de micro, mais je pense que ça marche, ça marche monsieur le président, madame la rapporteure générale et mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la rapporteure générale a rappelé qu'effectivement d'une part, le secteur des des grossistes répartiteurs a joué un rôle déterminant pendant la crise sanitaire et qu'il joue au quotidien un rôle déterminant pour acheminer les médicaments jusqu'au dernier kilomètre, c'est-à-dire jusqu'à la pharmacie et c'est la raison pour laquelle, comme l'a rappelé la rapporteure générale, un certain nombre de gestes ont été réalisées par le gouvernement à destination de ce secteur, ils ont été rappelés, la modification des marges réglementées, la baisse du taux de 1 virgule 75 à 1 virgule 5 % avec un effet rétroactif pour l'année 2021 et puis enfin l'introduction d'un forfait spécifique à la distribution des produits froids. L'ensemble de ces mesures mises Boutabout constitue un effort de 90 millions d'euros. La la mesure qui est proposée par la version la maximaliste des amendements de cette discussion commune qui consiste, consiste à faire baisser le taux de 1 virgule 5 % à 1 % représenterait un coût de 70 millions d'euros, il nous paraît pas nécessaire de à ce stade, en tout cas, d'aller au-delà des 90 millions d'euros déjà consentis, c'est la raison pour laquelle la vie est est défavorable sur cette série d'amendements dirais une une une assurance qui qui vous est donnée par le gouvernement qu'une attention toute particulière est accordée à ce secteur pour s'assurer qu'effectivement ces marges lui permettent d'assurer son service essentiel au bon fonctionnement de notre système de santé. Merci Monsieur Beulin. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègue le sujet que vient d'aborder notre collègue Chassaing et est essentiel pour nous, élus des territoires. Pour ça qu'il faut éviter de trop dézingué le prix du médicament tout à l'heure notre collègue Folio a bien fait d'insister sur le fait que, historiquement, avant l'arrivée des des génériques à peu près 15 % de la marge du prix était consacré à la recherche, c'est-à-dire qu'on travaille actuellement sur les médicaments qui sortiront en 2032 2035. Vous imaginez, il a fallu, je prends un exemple sur lequel j'ai vu l'occasion étudiants de suivre le a mis douze entre ces essais thérapeutiques et l'utilisation chez le patient, et là on parle de la répartition et Daniel Chassain, à raison de l'évoquer, parce que la répartition est aussi en danger si on. Des hein que je reprends cette expression, le prix du médicament parce que la répartition se rémunère sur le médicament et aujourd'hui on assiste à un phénomène simple : le rachat de groupe et le rachat de répartiteur, pas plus tard que la semaine dernière un grand groupe européen a racheté un groupe français l'OCP, je le cite parce que ceux qui connaissent le milieu, savent que c'est un groupe qui voilà, allez dans chaque pharmacie parfois en allongeant une tournée parfois pour une caisse et bien souvent, pour rendre plus service qu'autre chose, mais la disparition de ces répartiteurs par des grands groupes européens va remettre en cause ce système de répartition et demain matin, ils vont expliquer aux officines et donc derrière aux patients ben qu'y aura peut-être plus de livraisons par jour il y aura peut-être plus qu'une, puis qu'un jour il fera peut-être aller chercher les médicaments sur l'autoroute et donc défendent la répartition c'est défendent le patient et ses défendent le territoire merci monsieur le président. Merci, cher collègue Monsieur Savary. Hé bien, mais je je partage entièrement monsieur le Ministre, vous annoncez des chiffres et moi j'ai pas les mêmes chiffres,

franchement, c'est un secteur qui peut être en difficulté si on veut que le service se maintiennent, faut être attentif pourquoi. Hé ben demain côte il y aura plus qu'une boîte de médicaments, les délivrer dans un coin rural au fin fond de nos campagnes, ben ils n'iront pas parce que ça coûtera plus cher de faire la livraison que de la refuser, donc il y aura plus de service et quand on demande à nos personne d'être particulièrement attentif et de faire des efforts par rapport à cela et il faut aussi que parallèlement l'État montre l'exemple, par rapport à un secteur qui marche, qui a fait preuve, on a bien été content de les trouver, quand même, pour distribuer les vaccins parce que si on avait attendu que la stratégie logistique de santé publique France ben on n'était pas prêt d'en avoir, hein, parce qu'il y avait pas la même connaissance de terrain, alors c'est pas un procès d'intention que je leur fais, ils ont découvert, après il s'ils sont bien mis, hein, il y a pas de problème, mais simplement à la distribution en milieu rural notamment et et sur toutes les les pharmacies de France, ben ça c'est bien fait au départ par les distributeurs, donc soyons attentifs à cela, c'est la raison pour laquelle j'invite mes collègues ah suivent l'amendement que nous avons proposé de façon similaire Chassaing et moi-même. Si cher collègue, donc je mais aux voix les trois amendements identiques 266 527017 qui ont reçu 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés et donc ils font tomber les 3 autres 267 359018. Nous passons 794 Madame Cohen. Donc ça va pas du tout dans le sens de ce qui a été voté, vous vous en doutez, mais c'est ça le débat suite aux travaux menés dans le cadre du rapport d'information sur les médicaments, mes chers collègues, je vous rappelle que des pratiques abusives ont pu être mises en en lumière certains grossissent répartiteur répartiteur pardon dix short-liners attirés par la rentabilité du marché, notamment par le biais d'exportations parallèles développent leur activité sans respecter leurs obligations, parmi celles-ci, les grossistes répartiteurs doivent notamment disposer d'une collection suffisante de médicaments qui nécessite des capacités de stockage ainsi que celle de livrer les officines dans les 24 heures ses obligations entraîne un coût pour le fonctionnement des grossistes répartiteurs, mais celles-ci sont indispensables pour assurer un approvisionnement adéquate aux patients le non-respect de ses obligations peu compliqué, la traçabilité et entraîné des pénuries, car certains short-liners achète des médicaments à moindre coût en France pour le pour les revendent dans d'autres pays européens ainsi afin d'encadrer et dissuader dissuader, pardon, les pratiques abusives de certains grossistes répartiteurs, nous proposons cet amendement prévoyant une majoration du chiffre d'affaires, pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque les ces derniers ne respectent pas leur obligation de service public, je vous remercie. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes chers collègues, d'abord faire peut-être la distinction entre l'activité de grossiste répartiteur et l'activité de short Line, qui sont 2 activités différentes qui effectivement ne répondent pas aux mêmes obligations certains grossistes près répartiteur effectivement peuvent avoir une activité de short-liners mais qui est séparée, ceci étant un grossiste répartiteur qui ne respecterait pas ses obligations de service public peut déjà être sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende ne sont pas souhaitables de prévoir un second régime de sanctions en majorant dans ce cas, le chiffre d'affaires, pris en compte aussi de la contribution conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ouais, mais je pense qu'il faut faire effectivement le la différence, hé bien la différence entre les 2 activités, Même avis défavorable, donc je mets aux voix l'amendement 794 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'article 9 terre avec une prise de parole de Madame Cohen. L'Assemblée nationale a adopté un amendement demandant un rapport au gouvernement sur l'état et les perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, nous savons par avance le sort réservé par le Sénat, aux demandes de rapport, a fortiori dans une loi de financement de la Sécurité sociale, mais je vais donc profiter de cet article pour intervenir à nouveau sur la nécessité de doter notre pays d'un pôle public du médicament et des produits de santé souverainetés d'autres souveraineté sanitaire la pandémie de Covid et les ruptures de stock de médicaments révèle chaque jour davantage l'urgence de rétablir une industrie public du médicament capable de produire dans notre pays et de fournir l'ensemble des médicaments d'intérêt thérapeutique majeure, les politiques publiques en matière pharmaceutique ont accompagné les délocalisations de la production en Asie du Sud-Est, notamment, et aujourd'hui les firmes pharmaceutiques comme Sanofi font du chantage à l'emploi pour ouvrir des lignes de production, nous attendons d'ailleurs toujours la production du vaccin de Sanofi contre la Covid 19 après avoir bénéficié de milliards d'euros de crédit impôt recherche et supprimer des milliers d'emplois dans mon département, le Val de Marne, cette entreprise se comporte comme Amazon et Hubert avec un mépris des règles fiscales, sociales et environnementales, nous aimerions connaître, Monsieur le Ministre votre projet pour permettre à nos concitoyennes et concitoyens qui subissent des. Pénurie de médicaments et doivent modifier leur traitement, faute de disponibilité de leurs traitements habituels donc savoir comment hé bien, on peut avoir une intervention importante souveraine parce que pour nous, le médicament c'est pas une marchandise, c'est un bien commun. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, comme l'a pratiquement annoncé Laurence Cohen c'est un amendement de suppression parce que parce que proposition d'un d'un rapport donc effectivement, reconnaissez-le et on peut tout s'en être témoin, les rapports sont rarement transmis au Parlement, néanmoins, compte tenu de, de l'enjeu parce que le montant OM est devenu un vrai dispositif fiscal et je peux reprendre les propos d'Alain Milon et notre collègue Folio tout à l'heure, en tout cas c'est comme ça qu'il est ressenti et qu'il est vécu par le secteur du médicament, donc je ne doute pas que vous allez travailler sur cette clause de sauvegarde, M. Le monde le fonctionnement a profondément évolué ces dernières années le fonctionnement il est revu chaque année, ce qui en fait un mécanisme instable, sa nature a progressivement évolué de dispositif de dernier recours, la clause est devenu un mécanisme fiscal déclenché presque chaque année depuis 2015, surtout de l'incidence de la clause explose, si elle a généré des remises de l'ordre de 34 millions d'euros en 2018 126 millions d'euros en 2019, elle pourrait générer 750 millions d'euros en 2021, d'après les entretiens que nous avons eu avec le l'aime comme avec le ce PS. Les industriels craignent que son montant soit encore supérieur en 2000 22 et en 2023 6 7 7 un dispositif fiscal alors effectivement, je vous invite à en discuter avec les entreprises du médicament avec de la concertation à faire d'un dispositif qui soit équilibrée stabiliser qui donne de la lisibilité aux entreprises et surtout qui soient adaptés à la taille des entreprises parce que ce que disait notre collègue Folio tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui la France est en queue de peloton au niveau européen en termes d'attractivité à cause de sa fiscalité, c'est une réalité, vous pouvez le vérifier, je suis sûr que vous le savez, donc, alors que la l'haleine, l'année dernière à la même époque, on souhaitait voir, revoir les entreprises du médicament venir s'installer en France à défaut en Europe pour être retrouvé un peu d'indépendance sanitaire la ficelle qui s'y applique au contraire est complètement dissuasif. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, peut-être d'abord un, un élément de réponse pour Madame Cohen et pour la la rapporteure générale, simplement pour dire que, une nouvelle fois la la souveraineté industrielle en santé, elle ne se joue pas uniquement avec la clause de sauvegarde et avec les discussions autour des prix, je vous ai tout à l'heure si. Les les les. Crédits inscrits au titre de France 2030, mais je voudrais vous donner un exemple, beaucoup plus précis encore, qui concerne le le territoire de de l'Isère, puisque vous savez que dans le cadre du plan de relance 100 millions d'euros ont été consacrés à l'installation de séquences qui va permettre de re fabriquer du paracétamol en France et de fournir ainsi Sanofi et UPSA de manière souveraine et donc on on va en faire bénéficier le territoire évidemment de de l'Isère, mais également le territoire du Lot-et-Garonne ou UPSA à une implantation historique très important donc cette souveraineté industrielle en santé, elle se joue aussi dans une politique industrielle offensive et directe par le biais des subventions qu'on a pu voir dans le cadre du plan de relance, mais également dans le cadre de France 2030, ensuite, s'agissant du rapport, je crois que les débats que nous avons eu sur sur ces différents articles démontre que la la régulation est insatisfaisante les les mêmes débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale où les députés comme les sénateurs se sont aperçus ou le savent, déjà bien depuis longtemps que les mécanismes que nous avons de régulation, et singulièrement le rôle de plus en plus important qui est joué par la la clause de sauvegarde sont insatisfaisants et c'est la raison pour laquelle les députés ont ont souhaité que le gouvernement puisse sera remettre un rapport, alors il est, il est un peu différent des rapports remis par le gouvernement, habituellement puisque des personnalités qualifiées, vont être désignés pour superviser la rédaction de ce rapport et le je crois que le gouvernement en 1er lieu à tout à fait besoin de ce travail pour avancer sur cette question là, mais que le Parlement aussi bénéficiera de de l'éclairage de ce rapport et c'est la raison pour laquelle, même si c'est peut-être un peu moins dans les habitudes du Sénat que dans celle de de l'Assemblée nationale que de solliciter des rapports du gouvernement même si quand on, quand on s'acharne, on a, on finit toujours par les par les obtenir, je, je vous invite mesdames et messieurs les sénateurs à à ne pas adopter ce cet amendement de suppression et donc à valider le l'option des députés qui consiste à obtenir, voilà un un rapport et des éléments pour objectiver le le problème, essayer de trouver une solution durable. Non. Merci, monsieur le Ministre, non Monsieur Savary. Oui, rapidement, Monsieur le Ministre je là je vous trouvez sincère dans vos propos mais je commence à douter de la sincérité là parce que quand on rencontre les parce que lors des auditions, on a rencontré l'aime, c'est quand même le le syndicat qui regroupe toutes les les industries du médicament ils ont pas tout à fait le même le le même discours que ce que vous nous tenez, tout ne va pas aussi bien, j'ai l'impression d'entendre encore à un des membres, dire que ils étaient désolés, quand ils avaient découvert ce PLFSS donc quelque part, la confiance peut parfois être mise à mal, me semble-t-il, donc tout ne va pas aussi bien que ce que vous nous dites, et puis vous avez inventé l'article 9 terre alors moi je me suis dit il y a quelque chose qui m'a échappé, quoi, donc j'étais impatient de découvrir l'article 9 terre. C'est un rapport. Des rapports, on va proposer, combien cinquante soixante là parce que c'est une façon pour aborder un problème pouvoir en discuter, sinon on est soumis aux articles 40 45.

on vous fera plus confiance en prenant des engagements directement en vous entendant que nous proposer un rapport, c'est la raison pour laquelle, moi en tout cas je ne voterai pas le rapport et je suivrai la proposition de notre excellente rapporte. Puisque vous semblez apprécier les rapports, faites-nous un rapport, nous n'avons pas besoin pour cela de créer une clause dont la force obligatoire est nul, vous le savez d'ailleurs. Merci, chers collègue je mais aux voit cet amendement 41 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté et donc l'article 9 ter est supprimé, nous passons au titre de les conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale avec l'article 10 3 amendements identiques, le 720 Madame Poncet Monge. Merci monsieur le président, le présent amendement conteste la pertinence et le sens du transfert de la charge des indemnités post-natale de la CNAM à la CNAF si nous pouvons être favorable, quelques fois au principe de solidarité transversale entre les branches, sécurité sociale, conscient de plus de ce que l'imputation de certains cours relève de conventions ici entre santé de la mère ou politique familiale ce transfert de 2 milliards qu'il trouve sa justification première dans les excédents de la branche et d'abord contestable en regard des besoins non couverts de la branche famille, en effet, les mesures de la branche famille présente dans ce PLFSS aurait mérité d'être moins restrictive en regard de la lutte contre la pauvreté des familles et des femmes et des enfants ou pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, car effectivement elle se limite aux familles monoparentales, alors que la pauvreté des enfants concerne bien plus de familles, même si des familles monoparentales sont plus impactées et aussi alors que la prolongation jusqu'à 12 ans de la CSG permettrait de mieux lutter contre le temps partiel subi souvent de la femme, des couples modestes comme des couples tout pareillement aux enfants, aux parents d'enfants en situation de handicap aux parents en situation de handicap, eux-mêmes, de surcroît, rien n'empêche de prévoir la revalorisation du congé parental, le fameux prépare dont le forfait ridicule rédu du curieusement bah n'a pas permis au 2ème par et en fait le deuxième parents c'est le père d'en bénéficier, générant une économie de près d'un milliard à la CNAF, il est des excédents non vertueux, monsieur le Ministre, qui assigne encore de facto les femmes au travail reproductif, cet amendement vise donc à souligner l'urgence de revaloriser les prestations de la branche famille pour une utilisation conforme aux missions de la branche et non, c'est pour cela que nous contestons ce transfert, je vous remercie. Merci, mes chers collègues de m'aider à m'y retrouver, mais vous inquiétez pas, je suis le débat, donc c'est effectivement. un amendement qui est identique pour les raisons qui ont été développés, je pense qui qui nous rassemble, c'est la la la suppression donc que nous demandons-nous également de cette. C'est cher collègue le 1043 madame Lubin. Défendu. Si Madame la rapporteure. Oui, alors je vais peut-être défendent mon amendement, si vous le voulez bien monsieur le président, c'est ça.

moi je présenterai ensemble ensuite un amendement qui fait comment, état d'une partie simplement de suppressions mais qui garde cependant une disposition. Qui souhaite conserver les précisions qu'il apporte au sujet des modalités de compensation de la réduction de cotisations sociales des travailleurs indépendants au moyen de la TVA, c'est quelque chose qui a été votée cet été et donc ça, il ne faut pas l'enlever de l'article, donc c'est un avis de défavorable à vos amendements. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le le président, mesdames et messieurs les les sénateurs un avis défavorable du Gouvernement sur les amendements de suppression de l'article qui vient transférer le le financement des années des indemnités journalières maternité post-natal à la branche famille, c'est une recommandation qui a été faite par la Cour des comptes et qui ne vient pas entamé la détermination du gouvernement s'agissant de la politique familiale, puisque ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale comporte notamment la Linea réalisation c'est-à-dire légalisation du reste à charge pour l'accueil des des des jeunes enfants qui d'ailleurs adresse une partie des préoccupations exprimées par les auteurs des amendements que qui viennent d'être présentés, s'agissant des familles les plus modestes voilà, mais en tout cas un avis défavorable sur sur ces amendements de suppression. Merci monsieur Oui c'est, explications de vote, les avis ont été donnés. puisqu'il me semble important qu'en effet, ces 2 milliards soit utilisé au niveau de la Caisse d'allocations familiales et non pas par ailleurs, je voudrais vous rappeler, Monsieur le Ministre quand même que sous la mandature de Monsieur Hollande la Modus il y a eu, a été mis en place la modulation des allocations familiales l'effet depuis 2014 de cette modulation des des questions familiales, c'est une moindre recette pour les familles de près de 4 milliards, ce qui n'est pas rien quand même, il a été mis en place aussi la suppression du complément de libre choix d'activité majoré, il a été mis en place la la modulation de la fameuse page là l'allocation de base, la prestation d'accueil du jeune enfant et il a été mis en place l'alignement du montant du plafond de l'allocation de base sur le complément familial les excédents de la de la branche famille qu'on a actuellement, aurait pu servir à compenser ses déficits aux familles et à remettre en place une vraie politique de natalité, plutôt que de remettre 2 milliards sur la caisse de de santé il y a entendu de sécurité sociale branche santé de milliards qui de toute façon ne rééquilibre ont pas malheureusement les comptes de cette caisse puisque, avec ses 2 milliards en plus, on a quand même un déficit de près de 7 milliards prévus, je vous rappelle que pour 2022, c'était 6 milliards prévus et qu'on est à près de 13. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi aussi, je voterai l'amendement il a pas pu encore être expliqué mais on doit bien expliqué puisque le le débat est ouvert en tant que rapporteur de la branche famille des raisons pour laquelle il faut revenir sur ce ce transfert, parce que bien évidemment il y a quelques lueurs, vous les avez exposés Monsieur le Ministre, les évolutions sur la CMG pour les les familles monoparentales, l'augmentation de 50 % c'est vrai que ce sont des lueurs mais il y a quand même peu d'ambition en matière de politique familiale de la part du gouvernement, alors qu'on a une branche qui est bénéficiaire qui excédentaire de 3 5 milliards qui d'ailleurs de des des effets des des mesures ce cet excédent diminué à 500 millions dans 2 ou 3 ans, ce qui fait que, au moment où on veut afficher une ambition peut être revenir sur la modulation peut être créer un service public de la petite enfance, hé bien, je crains que il n'y aura plus d'argent pour assumer cette cette ambition, alors même que la création de places de crèches est indispensable, on sait que c'est ça, ça c'est une évidence en termes d'égalité femme c'est aussi à un des freins au retour à l'emploi avec ma collègue, Frédérique Puissat, on travaille sur ce sujet, on voit bien que, en matière de retour à l'emploi, la question des places de crèche et est une question tout à fait essentiel et au moment où on va devoir afficher d'ambition, hé bien on aura plus de moyens, je trouve que il y a pour le moins une un paradoxe et même je dirais une contradiction, je vous remercie. Si cher collègue, donc oui, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, simplement en complément de ce que monsieur le sénateur, et nos vient de vient d'évoquer, rappeler qu'une fois ce transfert réalisé si le le le le Parlement l'gré qu'une fois le le l'égalisation du complément mode de garde acté, c'est 2 6 milliards d'euros qui qui serait transféré sur la branche famille qui resterait néanmoins excédentaire à hauteur de 700 millions d'euros, et par ailleurs s'agissant de la du financement qui est transféré, rappeler que c'est une aussi une mise en cohérence avec la la façon dont le congé paternité le a été inscrit, puisqu'il est financé lui aussi par la branche famille et qu'il s'agit bien là de transfert de transférer le le financement non pas

en dépit, si je puis dire de ces transferts de 2 milliards plus 600 millions la branche reste excédentaire à hauteur de 700 millions d'euros et qu'il y a là une mise en cohérence avec les décisions qui ont été prises, s'agissant du congé paternité. Merci, monsieur le Ministre, oui madame la présidente. Oui, j'entends ce que vous dites cette comparaison avec le congé paternité, c'est pas du tout la même chose : un congé post-natal c'est c'est la femme qui accouche et c'est un problème de santé il y a un problème sanitaire et c'est pas un problème simplement de ce qui se passe après un accouchement, pour que la femme reste chez elle sert, ce qui est bien pour s'occuper de l'enfant mais aussi quand même une notion sanitaire, donc c'est pour ça que nous souhaitons que ça reste à la branche maladie.

Qui s'abstient, ils ne sont pas adopté l'amendement 42 la commission du coup madame la rapporteure. Oui, alors du coup je, je dirais que vous avez anticiper les choses mais, chers collègues, mais l'amendement que je propose, justement, s'oppose à ce transfert de 2 milliards d'euros de charges sur la branche famille, pourquoi, parce que, comme l'a dit, certaines personnes ici déjà, hé bien, par rapport à la politique ambitieuse que veut mener aussi la CNAF, hé bien, là, elle se retrouverait avec finalement un montant de ressources, ce qui serait tout de même assez faible, je voudrais dire aussi que la présidente, madame, Isabelle Sancerni a eu l'occasion d'envoyer aux uns et aux autres, le courrier du conseil d'administration qui montre bien que s'ils sont favorables, mesures de ce Plfss en matière de petite enfance, il trouve que ce n'est pas normal non plus que de prendre 2 milliards d'euros parce que, en fait, cette branche serait aujourd'hui excédentaire il trouve même aujourd'hui que leur situation est fragile, ils disent même que le service aux familles a dégradé ce qu'il souhaite, c'est avoir les moyens de mettre en oeuvre la prochaine code qui est actuellement en négociation, donc il faut bien voir là que les difficultés elles seront importantes, il faudra vraiment prendre en compte l'ensemble des propositions qui ont été données par mes collègues et qu'il faut donc laisser ces 2 milliards d'euros sur la branche famille, parce que c'est nécessaire, la branche famille, la CNAF le dit, mais nous, nous le disons aussi depuis de nombreuses années, la politique familiale en France n'est pas assez ambitieuse, il faut y mettre les moyens et ce n'est pas en ponctionnant en faisant ce ce ce transfert finalement que on on va avoir les moyens de cette ambition, donc c'est un amendement de suppression de cette partie là de l'amendement. Oui, à nouveau, simplement rappeler que ce transfert n'entament pas la détermination du gouvernement à mener une politique familiale ambitieuse non le congé le le doublement du congé paternité, ça n'est pas tout à fait rien, c'est quand même quelque chose en matière de politique familiale, légalisation du complément de mode de garde, c'est également quelque chose d'intéressant reste excédentaire, ce qui lui permettra de mener des des des politiques en en en soutien aux familles le le sénateur et nous a rappelé tout à l'heure qui a cette ambition cet horizon d'avoir un service public de la de la petite enfance, nous ne renonçons pas à cet horizon, même si c'est évidemment un projet suis structurant qu'il nous faudra sans doute quelques quelques années beaucoup de travail pour y parvenir mais je, je, j'insiste pour dire que ce transfert n'entame pas la possibilité pour la la la caisse et pour le pays de se de 2 poursuivent la construction de cette politique familiale ambitieuse. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur Savary. Ouais, non mais Monsieur le Ministre, une embrouille tout ça hein. Parce que si il y a des branches notre sécurité sociale, c'est bien pour montrer une certaine politique il y a une politique de la santé et il y a une politique familiale une politique familiale, c'est pas forcément une politique sociale, ces différences sont des critères autre où on veut favoriser la natalité ou dose d'autres choses, si vous voulez, si vous voulez donner de moins de charges à la branche famille, vous lui mettez moins de recettes, c'est elle a moins de responsabilité que il y a des modifications au niveau des recettes pour faire la politique de la branche, ça peut se comprendre, mais que l'on ponctionne 2 milliards sur la branche famille pour un remettre à la branche maladie, un milliard sur la branche AT-MP et il y a qu'à supprimer les branches Monsieur le Ministre, ce sera beaucoup plus facile, tout ça c'est des embrouilles, on a eu la discussion hier avec le ministre de la santé qui fait des annonces 400 millions d'euros extraordinaire, sauf qu'il y a pas de recettes supplémentaires, donc c'est des fonds qui sont affectés différemment, donc rien ne change, ce sont des annonces mais concrètement l'argent qui devait à aller l'hôpital hé ben il va aller à l'hôpital, il y en a pas plus d'argent qui ira à l'hôpital, et là c'est pareil, il y a pas plus d'argent qui ont chez familles. C'est la raison pour laquelle on s'oppose à ce transfert, donc soyons attentifs à cela, c'est le maintien des branches de notre sécurité sociale, surtout quand on en fait une de plus, quoi, parce que maintenant il y a la branche autonomie alors si on prend les fonctions de la pour remettre à l'autre, on a rien gagné, tout ça c'est des jeux de tuyauterie budgétaire qui ne répondent pas aux préoccupations de nos concitoyens.

je voudrais dire que la dernière, je l'ai dit dans mon intervention, la dernière, la réforme de ah prépare un qui a cantonné le congé parental en 2 ans maximum pour un parent et un an pour l'autre en mettant une forme une somme forfaitaire complètement ridicule, vous saviez déjà parce que, paraît-il, c'était déjà

réforme la contre-réforme de la prépare, vous voyez nous mettrait mettrait la peur, la, la branche famille en déficit puisque vous dites qu'il va y avoir 800 millions et là on a économisé un milliard 100 donc là, vous voyez bien que que c'est pas raisonnable de dire que, à partir du moment où il reste encore quelques miettes, on ne porte pas atteinte à une politique familiale dynamique et celle qui permettrait notamment au père parce que c'est souvent le père de prendre l'année de 2 prépare de 2 prépare qui ne prend pas à cause de cette somme ridicule monsieur ce président ce ministre je j'entends bien ce que vous dites par rapport aux excédents de la branche famille mais je rejoins à ce qu'il a dit, René-Paul Savary lorsque, en 1945 les branches ont été créées, elles ont été créées avec des définitions extrêmement précises et des missions extrêmement précises, j'ai dit hier dans mon intervention ont ponctionné déjà un peu trop allègrement un peu trop facilement la branche AT-MP depuis des années et suivant suivant différents gouvernements mais ce que l'on constate que lorsque l'on regarde la natalité dans notre pays,

on a une diminution progressive de la natalité de la natalité, il faut donc peut-être faire un effort sur la politique familiale et la politique de natalité pour essayer de remonter cette natalité avant qu'on se retrouve dans la même situation que l'Allemagne d'être obligé de faire venir une population étrangère pour faire le travail qu'il ne peut plus être fait part à l'absence de français. Merci, cher collègue Madame pour ce. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, moi aussi, je pense qu'il faut garder ses branches avec ses missions, c'est d'ailleurs ça le budget de la de la sécurité sociale, c'est les branches et ses missions et les missions qui sont dévolues à chaque politique monsieur le ministre, enfin moi j'ai quand même un souci alors je sais bien, on n'est pas très intelligent, on est parfois, mais vous êtes en train de nous expliquer que vous allez enlever. 2 milliards de la branche famille et que vous gardez les mêmes ambitions. Mais enfin, on marche sur une autre moins c'est moins comment voulez-vous garder les mêmes ambitions si vous enlevez de milliers de la branche famille, vous nous prenez pour des, enfin bref, voilà un an, mais quand on enlève 2 milliards on enlève 2 milliards enfin vous m'excuser comme vous voulez, les mêmes ambitions mais qu'est-ce que ça veut dire alors qu'il a tant à faire sur la branche famille, il y a tant à faire, enfin voilà, expliquez-moi un peu, voilà comment vous voyez les choses à voir les mêmes ambitions, avec 2 milliards en moins, expliquez moi les choses. Peut être là aussi pour mettre un tout petit peu les choses en perspective, n'allons pas dire que la la France n'a pas de politique familiale. Les dépenses de la branche famille, c'est quand même 50 milliards d'euros pour 2022, et c'est plus 5 milliards d'euros si nous adoptions si vous adoptiez, si le Parlement a adopté le texte que nous sommes en train de discuter, c'est plus 5 milliards d'euros sur une base de 50 milliards d'euros, n'allons pas dire que nous n'avons pas de politique familiale ensuite qu'il y ait des projets qui mérite d'être conduit à l'avenir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le avec comme horizon le service public de la petite enfance, qu'il ne peut qu'il ait une vraie et grande politique familiale et la branche famille conserve des capacités d'action, j'entends les arguments qui ont été livrés, mais la branche famille conservent une capacité d'action et quant aux transferts inter-branches,

ça a existé parce que la sécurité sociale et permanente, mais les besoins de chaque branche évolue et donc nous avons là un transfert qui une nouvelle fois n'entame pas le la capacité d'action de la branche famille, dans le cas d'une politique familiale qui dans notre pays reste ambitieuse, comme en témoigne le chiffre, le chiffre associé à ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, plus 50 plus 5 milliards, on passe de 50 milliards à 55 milliards pour 2020.

C'est une suppression du principe de non-compensation à la sécurité sociale, du coup, de la prime de partage de la valeur, c'est donc ce ce c'est les articles 21 et 22 qui sont concernés et qui sont supprimés par cet amendement.

la compensation des exonérations de cotisations appliquées à la prime pour le partage de la valeur, celle-ci représente pourtant une perte de recettes massives pour les comptes de la Sécurité sociale en effet au 1er trimestre 2019, le salaire moyen par tête a augmenté de 2 7 % sur un an, soit la plus forte augmentation depuis 9 ans, selon l'Insee. Mais si on exclu de la masse salariale, les 2 2 milliards d'euros perçus par les salariés au titre de la prime pas hé ben ce salaire moyen par tête n'aurait progressé que de 1,3 % sur un an, la progression serait ainsi inférieure à celle des trimestres précédents ou suivants, ce qui conforte quand même la forte présomption d'importants effets d'aubaine des incitant les gens, les employeurs à augmenter les salaires de leurs ça employé et qui accorde en substitution des primes évitant, impôts et cotisations, nous ajoutons que cette prime est loin de toucher de manière uniforme égalitaire, les travailleurs, vous le savez, je vous renvoie aux statistiques, en conséquence, considérant que ce n'est pas aux comptes de la Sécurité sociale, de financer une mesure en plus qui des incite à l'augmentation des salaires, sur lequel, quand même, la Sécu puise ses recettes, cet amendement vise à maintenir la compensation par l'État du manque à gagner pour les comptes de la Sécurité sociale que représente la prime pour la pour la pour cette compensation avait en outre été adoptée par le Parlement cet été à l'occasion de l'adoption de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, je terminerai en disant qu'il y a une politique délibérée et je dis bien délibérée d'exonérations non compensées d'assiettes, elles sont totalement non compensée pour conduire à un constat de caisses vides ou de déficit, justifiant la nécessité, ensuite, de baisser les dépenses publiques.

partage de la valeur depuis le 1er juillet 2022, les employeurs peur verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et cotisations et contributions sociales dans la limite de 3000 euros et jusqu'à 6000 euros pour les entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation lors de l'examen de la loi, pouvoir d'achat, notre collègue député communiste. Pierre Dharréville avait d'ailleurs fait adopter un amendement précisant que la prime de partage de la valeur sûre et intégralement pris en charge par l'État, conformément à l'article L 131 7 du code de la sécurité sociale, notre collègue puis ça avait estimé selon la page trente-deux du rapport sur la loi que l'article L 111 je 3 du code de la sécurité sociale de valeur organique prévoit déjà la compensation par l'état de toute mesure de diminution des recettes de la Sécurité sociale adopté en dehors d'une loi de financement de la Sécurité sociale de plus jusqu'à présent, le gouvernement a toujours affirmé que les prime exceptionnelle, de pouvoir d'achat n'aurait pas été versé en l'absence de dispositions législatives et n'avait donc pas de coup Direct pour la sécurité sociale et ajouté, je cite toujours, il a encore adopté la même approche dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi pour ces 2 raisons, cet amendement pour sympathique qu'il soit dans son principe n'aura pas d'effets opérationnels dès lors, cette disposition est une honte pour le gouvernement qui ne respectent ni les parlementaires ni la démocratie, et ni les assurés sociaux qui vont payer eux-mêmes la prime de partage de la valeur, désormais il n'y a ni partage ni valeur dans ce gouvernement,

qu'on appelle aussi parfois la prime Macron enfin la paix pas puisque elle a été conçue pour ne pas se substituer à du salaire ou à toutes vos autre forme de rémunération si nous acceptions ou si nous donnions un avis favorable à un amendement qui vise à compenser la prime la la prime paie pas, cela voudrait dire que nous acceptons le principe selon lequel cette prime se substituent à des modes de rémunération et comme nous ne l'acceptons pas comme cette dispositif n'a pas été conçu pour cela l'avis sera défavorable, en réaction au au commentaires qui ont été faits, s'agissant en général de la compensation par l'état de la sécurité sociale que d'une part, il était sans doute un peu exagéré de dire que, qu'elle n'existe pas puisque pour l'année 2022, ce sont 64 milliards d'euros qui vont être compensée de l'État au à la sécurité sociale et que c'est en croissance puisque pour 2023 si le Parlement a adopté ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ce serait 68 milliards d'euros, dont 4 milliards d'euros supplémentaires qui seraient compensées de l'État vers la sécurité sociale. Merci, chers collègue dont je mais on voit ces trois amendements identiques le 43 726 833 avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés je mais aux voix, l'article 10 ce qui est pour l'article 10. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté après cet article 10 l'amendement 1065 madame Meunier. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, hier soir nous avons débattu de l'instauration d'une redevance solidaire assise sur les revenus des Epad privé à but lucratif au bénéfice de la branche autonomie c'est une proposition, un amendement qui a été rejeté et toujours dans le même optique de trouver des moyens supplémentaires pour la branche autonomie, nous vous proposons ce soir un amendement qui crée une contribution de 1 pour 100 assis sur les revenus des capitaux mobiliers pour financer la 5ème, branche de la Sécurité sociale, on le sait, la 5ème, branche la branche autonomie a été créée, mais sans financement pérenne on sait aussi les besoins dans ce domaine, le rapport Libault de 2022, mais aussi le rapport que nous avons commis avec Bernard Bonne biais 2019 fait état d'un besoin de financement annuel, à hauteur de 6 milliards à partir de 2024 demain mais de 9 milliards à partir de 2030 concernant l'autonomie 2030, mes chers collègues, ça nous parle parce que nous y serons alors cet amendement donc propose une contribution assis sur les revenus des capitaux, c'est-à-dire les dividendes, les obligations, les bons de capitalisation, émis en en France et hors de France, le rendement de cette contribution serait de un milliard 500 millions donc le compte n'y est pas, mais c'est une première Pierre, un abondement de cette branche qui servait à s'occuper de nos aïeux de nos parents et peut-être aussi de nous dans les établissements mais aussi à domicile. Si cher collègue Madame la rapporteure. Oui, j'entends bien la préoccupation de notre collègue que nous partageons, mais en réalité, l'assiette de la contribution que vous créez une contribution de solidarité, hé bien, Le lien entre cette assiette de contribution et surtout le risque financé est assez mince et donc je pense que on on ne peut pas donner un avis favorable à cette proposition, j'ajouterai que pour financer la branche autonomie à partir de 2024 il y aura une fraction de la CSG, ça pourra en tout cas en partie compensé les les besoins que nous aurons sur cette branche autonomie c'est un avis défavorable.

c'est une proposition intéressante, alors nous n'allons pas voter au niveau de, de, de groupes et j'explique pourquoi, c'est parce que depuis le départ, nous sommes contre la 5ème, branche puisque nous considérons que le la, la, le vieillissement n'est pas un risque supplémentaire mais fait partie de la vie quand on on hé bien on vieillit et on meurt, c'est comme ça, donc il y a pas besoin de créer une 5ème, branche. Nous sommes minoritaires sur cette sur ce positionnement mais, donc nous ne pouvons pas voter un financement d'une branche. Pour laquelle nous sommes en désaccord, donc voilà pourquoi nous ne voterons pas cet cet amendement. Merci monsieur le président, moi je ne soutiens pas cet amendement parce que quelque part, c'est créer une taxe supplémentaire, un impôt supplémentaire, on le met sur cette thématique là mais on pourra le mettre finalement de de de capital, donc je crois que ce débat là d'être beaucoup plus globale et depuis le début, lorsqu'on évoque le financement de la ce qui est branche on on considère que nous n'avons pas de vision globale, il faut une stratégie, il faut des objectifs, il faut une connaissance des besoins et regard de planification des moyens financiers, donc là c'est un coup certains coups à milliards et demi qu'estimé même si il faut regarder de très près l'estimation, mais je crois que globalement on doit traiter les choses d'avec notre vision, et même si on a une tranche de la CSG, qui sera intégré dans les recettes à partir de l'année prochaine les on est juste sur un équilibre finalement de de la branche largement pas suffisant, donc il y a urgence finalement à bien définir la stratégie il y a urgence à trouver des moyens de financer pérenne et cette taxe qui est un coup quelque part un message n'est pas suffisant et moi j'invite vraiment le gouvernement à se poser pour réellement nous proposer une loi sur le tsunami avec une capacité financière pérenne et dans la durée. Oui, ben moi je vais soutenir cet amendement parce que de toute façon, oui, mais c'était une des propositions du rapport au Liban, le rapport, il a quelques années, on va différer jusqu'à quand, là, on a 2 ans déjà, où on a un déficit,

moi je dirais que 5ème branche ou pas 5ème, branche en tout état de cause, si, si on n'en chasse, j'aime bien cette idée d'enchâsser dans l'assurance maladie, le risque de perte d'autonomie, il faut que l'assurance maladie change de nom et qu'elle devienne l'assurance santé.

où l'on voit des gens qui chantent Marchons, marchons et qui reste inexorablement sur place, dont on a voté une loi en 2020 et depuis, vraiment, on n'arrête pas de dire : voilà, il va y avoir la prestation autonomie, l'autonomie, c'est une grande priorité, le président de la République, il le dit avec infiniment d'éloquence, c'est vraiment nécessaire, nous allons le faire et on ne le fait pas, voilà, alors on peut critiquer toujours toutes les dispositions que l'on peut proposer de toute façon, mes chers collègues, ça coûtera et ça coûtera cher, mais c'est une question de dignité, nous savons qu'il faudra le faire qu'il faut le faire, donc Madame Menier a proposé quelque chose de concret, nous sommes très ouverts à toutes les propositions concrètes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rester, monsieur le président, avec une coquille éternellement vide, ce n'est pas respectueux et ce n'est pas sérieux. merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, évidemment je soutiendrai cet amendement comme l'a dit et ma collègue, comme plusieurs l'ont dit, nous avons voté la création d'une 5ème, branche en août 2020 nous sommes en novembre 2022, rien ne s'est passé quant au financement pérenne, comme cela est indiqué, on nous dit aujourd'hui que la fameuse grande loi tant attendu sur l'autonomie promise dans le 1er mandat du président de la République, hé bien, aujourd'hui, cette loi, c'est l'Arlésienne parce qu'on nous a même dit il me semble dans ces débats récents que ben non, finalement on pourra faire autrement pour organiser les choses autrement, sans obligatoirement débattre ou en tout cas mettre sur la table ce te loin si attendu alors aujourd'hui avec cet amendement, c'est une proposition bien sûr, on sait très bien que ça n'est pas suffisant le le ma collègue l'a réaffirmé : les besoins attendus sont bien supérieurs, mais c'est un début, c'est une proposition qui montre que, voilà, avec des actes concrets, hé bien, nous pourrions être en capacité de rassembler et demi d'euros chaque année, c'est un début, il faudra poursuivre en ce sens. Merci monsieur le président je je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame Cohen, mais avant je suis quand même reprendre ce qu'a dit Madame Ferré, parce que la loi autonomie pour ceux qui ont l'histoire monsieur sueur de de cette chambre la loi autonomie, c'est la dernière année du mandat de Monsieur Sarkozy, où on en a parlé, il a nommé ministre à l'époque, qui est devenu d'ailleurs, la présidente de la CNSA et un an c'était insuffisant pour mettre en place cette loi et je me souviens très bien,

Assommé par Madame Delaunay qui m'avait dit : moi, monsieur, vous, vous n'avez pas fait la loi, autonomie, moi je vais la faire il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 12 ans de ça, alors il faut avoir de la mémoire, on peut reprocher en effet au président Macron de ne pas l'avoir fait, mais d'autres avant lui ne l'ont pas fait non plus. ça, c'est le 1er point le 2ème point, nous avons voté une loi monsieur sueur c'est vrai mais on en fait, on a voté une coquille vide, on a voté une branche autonomie sans conseil d'administration et sans, sans voir comment on allait financer cette branche autonomie, je suis d'accord avec Laurence Cohen, c'est pas la branche autonomie, on n'aurait jamais dû l'appeler 5ème, branche, on aurait peut-être dû l'appeler branche autonomie et avant de créer la branche autonomie, on aurait certainement dû penser à la façon dont on aurait organisé cette branche autonomie la façon dont on aurait financé cette branche autonomie donc une grande loi de, une grande loi autonomie aurait dû venir rapidement, elle ne vient toujours pas, mais elle ne vient pas à la suite des hésitations de monsieur Sarkozy dans le cas de sa dernière année du mandat de Monsieur Hollande dans le cadre de ces 5 années de mandat et de monsieur Macron dans le cas de son 1er mandat. Merci Monsieur Chassaing. Si on peut rester sur l'amendement, ça serait bien. Monsieur le président, oui, mais je, je veux parler de, un petit peu de l'autonomie alors attendez, oui, mais je m'exprime, bon moi je voulais remonter au au dernier Ministre de Jacques Chirac qui s'appelle Philippe Bas et et et donc j'ai lu le rapport de Philippe Bas, qui est un très bon rapport et qui disait lorsque le GMP arrivera à 730 il faudrait qu'il y ait un employé pour un pensionnaire et on est toujours à 0 6 employé pour un pensionnaire, dont 0 3 soignants et il faudrait au moins monter à 0 5 soignant si on montait à 0 5 soignant, ça ferait 5 employes de plus paraît hé bien ça fait à peu près, disons 3 milliards mais bien sûr, entre 2020 et 2030, il y aura à peu près 200000 personnes dépendantes en plus et il faudra encore créer autre chose, donc j'attends, on attend Monsieur le Ministre, c'est vrai que cette branche autonomie soit financé, vous annoncez, vous avez annoncé le ministre autonomie a annoncé ce qu'avait dit le président de la République 50000 emplois il en faut 35000 dans les EPHAD et il faut d'urgence effectivement qu'il y ait un financement par la CSG, merci. Merci, cher collègue Monsieur Richard. Oui, merci Monsieur le Président, c'est le ministre, mes chers collègues, moi j'ai voté cet amendement, ça va être, c'est étonnant, mais je le voterai pour 2 raisons : la première raison c'est que

d'aider enfin moi je ne comprends pas ce ce ce discours et deuxièmement c'est une coquille vide, on le sait bien, ça a été dit sur ces bancs, plusieurs fois, il faut bien remplir cette coquille enfin franchement, si c'est un risque, il faut quelque part il y a porté quelques moyens, moi je considère cet amendement comme un amendement d'appel, c'est la raison pour laquelle, franchement je je vais le voter. Merci monsieur Mario. Oui, on peut se renvoyer pendant longtemps le passé, ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, là ce que l'on vous propose ce soir à partir de l'amendement de Madame Meunier, c'est une solution concrète donc qu'on l'a dit, ça a été dit, c'est peut-être pas parfait, mais on est face à la enfin au on a une population qui vieillit, la perte d'autonomie, ça va être quelque chose d'important dans les années à venir et la façon dont on ne traitera cette perte d'autonomie et à mon sens une prise en compte de l'humanité tout simplement hein de d'être humain par rapport à à ce risque qui est un risque, c'est même pas un risque, c'est une certitude qu'on saura un jour ou l'autre tous confrontés à la perte d'autonomie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président peut être 2 éléments en réaction à ce qui a été dit, premièrement pour dire que d'initiative parlementaire, la création de la 5ème, branche est évidemment une une excellente nouvelle et que oui le la perte d'autonomie est un risque à la fois pour la personne âgée, mais aussi pour la personne qui,

2. Dès la loi de financement de la Sécurité sociale de 2021 c'était 33 milliards d'euros, qui était inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale que nous sommes, vous êtes en train d'examiner ce sont 36 milliards d'euros qui qui sont eux-inscrit comme vous le savez, en 2024 nous aurons un cliquer de 2 milliards d'euros supplémentaires, si bien qu'en 2026 nous avons déjà une projection à 42 milliards d'euros pour cette coquille qui n'est. Pas complètement vide, si l'on peut dire, même si évidemment elle est perfectible, s'agissant d'une branche qui a été créé, d'initiative parlementaire, il y a 2 ans seulement. Merci, monsieur le Ministre, dont je mais aux voix l'amendement 1065 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je vais aux voix, l'article 11 qui est pour l'article 11 qui et contre qui s'abstient, il était adopté, après cet article trois amendements identiques, le 466 madame Portillo Fontan. Merci monsieur le président, mes chers collègues, cet amendement répond à une attente exprimée notamment par l'Association des maires de France, une demande plutôt légitime qui s'inscrit finalement une recherche de bon sens, il s'agit de la contribution sociale de solidarité des sociétés plus connu sous l'acronyme ces le Conseil d'analyse économique, estime d'ailleurs que cette cotisation est l'impôt le plus nocif à supprimer en priorité cette cotisation présentent plusieurs désavantages tout d'abord, elle pénalise le processus de production, ensuite elle pénalise l'exportation puisque réduire l'impact de la c'est trois sur leur compétitivité, il devient plus intéressant donc pour les entreprises françaises de s'approvisionner à l'étranger à l'étranger où cette taxe n'existe pas et puis surtout la suppression de la S coûterait moitié moins à l'état que la compensation de la CVAE, il est donc essentiel à mon sens, en tout cas de sauvegarder le lien entre les entreprises et leurs territoires d'implantation, c'est donc l'objet de mon amendement que je soumets à votre appréciation chers. Merci de 660 Madame Gatel identique. Merci, merci Monsieur le Président, là on peut se demander ce que vient faire cet amendement, sachant qu'il a un lien avec le PLFSS trois c'est une contribution qui financent la branche vieillesse, donc elle correspond à 3 milliards 600000 euros, mais il ne s'agit pas du tout d'exonérer les entreprises d'impôts vous savez qu'il est fortement question de supprimer la CVAE qui est un impôt économique payée par les entreprises, mais sur les territoires, et je pense avec d'autres, ma collègue l'a dit et des associations d'élus que supprimer la CVAE c'est un danger énorme pour plusieurs raisons : d'abord parce que je pense qu'il y a un principe qu'on aime ici au Sénat, qui décide paye et décidé de supprimer un impôt qui appartient au territoire, c'est un peu gênant, donc l'État ferait mieux de supprimer des impôts qui le concerne il pourra compenser, deuxièmement, il y a un lien entre les territoires et la CVAE qu'il faut savoir respecter et quand on de voix, on va devoir mettre en place, Lausanne les territoires vont devoir choisir entre l'implantation d'entreprises et l'habitat, et je pense que s'il a plus de ressources, les territoires ne choisiront pas l'impôt et juste pour vous dire que nous sommes des gens très responsables, produit de la c'est 3 S, c'est 3 milliards 6 d'euros alors que si l'État veut nous compenser et ce sera un minimum la CVAE ces 9 milliards 5 d'euros mais comme l'État compense déjà 2 milliards elle ça ne ferait que 7 milliards, donc voilà ma proposition d'amendement

Oui merci, cher collègue pour votre proposition l'effet économique des impôts, de production et probablement néfaste et et vous l'avez dit, comme le souligne d'ailleurs l'auteur du premier amendement qui été exposée telle est d'ailleurs la logique de la suppression de la CVAE et ça a été rapporté par la seconde oratrice cependant l'affectation de la c'est 3 S, je vous le rappelle, est indispensable à l'équilibre de la branche vieillesse et donc il me semble que c'est pas tellement opportun de la supprimer et en réalité est-ce que c'est au moment du PLFSS qu'on doit finalement mettre mettre en doute le meilleur véhicule pour comparer les mérites ou les effets nocifs des contributions en tout cas, là c'est trois S et de la CV je, je pense qu'effectivement la question peut se poser, mais la réalité c'est que nous avons besoin de 3 S pour la branche vieillesse et que là, c'est un avis défavorable de la commission. Monsieur le Ministre.

celui de supprimer la c'est 3 S : celui du supprimer la CVAE la CFE-c'est pas, c'est pas un choix qui se présentent à nous, cette année, c'est un choix que nous avons déjà fait il y a un ou 2 ans,

Là c'est 3 S était tentant, pourquoi, parce que elle, elle frappe le chiffre d'affaires, c'est-à-dire dans le compte de résultat, un niveau plus élevé que que la CVAE, elle a donc des effets de distorsion des effets de de des incitations plus plus important et par ailleurs, on peut la soupçonné d'être répercuté en cascade dans les chaînes de de production, elle est donc potentiellement un peu plus toxique. Pour les chaînes de production que ne l'est la CVAE. Mais la raison pour laquelle la CVAE a été retenu en définitive, c'est que, comme vous le savez, il y a d'ores et déjà un abattement de 19 millions d'euros pour la C3, si bien que lorsque vous supprimez la c'est 3 S en réalité vous favoriser les entreprises qui ont d'ores et déjà plus de 19 millions de d'euros de chiffre d'affaires,

vous amputer le le le financement de la branche vieillesse et, enfin, par rapport à la CVAE vous avez tendance à plutôt favoriser les services et notamment les services financiers, que l'industrie et c'est pour ces raisons-là, le choix de soutenir les PME les ETI et de donner un coup de pouce à l'industrie, que c'est la CVAE qui a été retenue, lorsque nous étions au moment de la relance et, dans le cadre du projet de loi de finances, mais comme vous l'avez dit, il est évidemment indispensable que si la CVAE et supprimer que les collectivités soient compenser et je sais qu'un certain nombre de débats ont eu lieu dans les 2 assemblées sur ce sujet. Merci, monsieur le Ministre. Défavorable sur ces amendements de suppression de la. Donc je vais se voit ces deux amendements 466 Madame Gatel. Gatel. Le ministre, vous avez raison, c'est une décision et un choix que le gouvernement a fait et ça lui appartient, mais je voudrais rassurer mon excellente collègue rapporteur, il ne s'agit pas de supprimer des recettes, il s'agit de dire que l'État pourra compenser cette recette sur la branche vieillesse comme l'État sera amené à compenser au territoire la CVAE voilà monsieur le mini, c'est un choix que vous avez fait droit, que je voudrais simplement dire et vous le savez très bien, parce que je vois que vous connaissez bien le dossier, que le Conseil d'analyse économique, a estimé, a déclaré en 2019 que là c'est 3 S était l'impôt le plus toxique parce que c'est un impôt qui pénalise la production et l'exportation, donc voilà, j'ai bien entendu mais je vous invite à poursuivre la méditation à laquelle on vous encourager,

et elle est restée, et donc moi je vais vous dire, c'est un débat que nous vous nous ne devrions pas avoir et ensuite moi je soutiens tout à fait le lien aussi entre les impôts et les territoires, c'est essentiel, c'est ce que vous avez déjà enlevé avec la taxe d'habitation.

Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés, nous passons à l'amendement 766 Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, actuellement, l'assurance maladie prend en charge 80 % des dépenses de consommation de soins et de biens médicaux mais la répartition de la dépense par type de soins très contrastées et démontre que les soins de ville représente la première dépenses pour les ménages selon l'adresse 89 % des personnes les plus pauvres ont une complémentaire santé contre 95 % en population générale, les retraités qui, eu égard à l'orage on les cotisations, les plus élevés, les personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques, qui ne peuvent pas travailler les chômeurs et les travailleurs indépendants qui doivent prendre une complémentaire santé individuelle au prix fort et non déductible des impôts face aux inégalités dans l'accès aux complémentaires santé dans les couvertures qu'elle propose ainsi qu'aux coûts pour les assurés sociaux et l'État nous portons le projet d'un remboursement des dépenses de santé à 100 % par la Sécurité sociale, cet amendement reprend une proposition de loi déposée par notre groupe en juin dernier, visant à restaurer une sécurité sociale solidaire avec la suppression des barrières financières et des dépassements d'honoraires, avec le remplacement de la notion de panier de soins par celle de soins prescrits avec l'extension des remboursements aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap, l'intégration de l'aide médicale d'État au régime général d'assurance maladie notre amendement propose donc de rétablir les cotisations du CICE pour assurer le financement intégral des dépenses de santé, par l'assurance maladie en renouant ainsi avec les principes originels de la création de la Sécurité sociale, le remboursement des dépenses de santé à 100 % par l'assurance maladie va entraîner une réorientation des mutuelles vers leur mission de prévention et de promotion de la santé en organisant et développement notamment les de santé et en assurant la gestion des établissements médicaux et médico-sociaux tels et le sens de notre amendement et je veux rassurer notre collègue André Reichardt, l'autonomie, pour nous, elle sera prise en charge par l'assurance maladie, tout simplement. Si Madame la rapporteure. on a déjà eu ce ce débat en commission, je pense que ma collègue ne sera pas étonné, je voudrais lui dire tout de toute façon, mon respect pour la vision constante et cohérente du groupe CRCE sur ce que devrait être le financement de la branche maladie, mais à plusieurs reprises, on lui a aussi indiqué combien de Eton opposé à ces propositions, c'est donc un avis défavorable de la commission. Oui ça simplement pour rappeler, merci Monsieur le Président, que ces allégements de de de charges ne sont pas tout à fait des des cadeaux qui ont été faits au aux entreprises, puisqu'ils ont permis en en stimulant les les créations d'emplois, de contribuer à au financement de la Sécurité sociale, nous avons connu dans les cinq des années qui viennent de s'écouler, une création nette de 1 1000000 d'emplois je précise au passage que ces employes ou que c'est les, les, les créations d'en d'emploi ont été particulièrement dynamiques dans les départements les plus pauvres de notre pays, ces 5 dernières années comme l'a dit la la rapporteure générale la l'intention est constante et elle est, elle est sans doute louable mais revenir sur ces allégements de de cotisations de de manière assez brutale, comme vous le proposez reviendrait à à inverser cette trajectoire qui a permis non seulement de créer de l'emploi et en finançant la protection sociale, mais aussi de permet des créations d'emplois et d'emplois industriels, tout particulièrement dans les départements les plus fragiles. Oui, c'est le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le CICE, c'était bon quand même quelque chose qui était bien parce que ça a permis aux entreprises d'avoir un petit peu de marge et ensuite je pense que c'était bien aussi de pouvoir diminuer les charges pourquoi diminuer les charges, mais par rapport aux autres pays parce qu'on est dans un pays européen et il y a une compétition et donc ça a permis effectivement à mon avis, enfin, enfin, quand on le lit, c'est ça, de créer des emplois tout à l'heure, je peux vous vouliez intervenir sur la CVAE parce que je pense que il faut essayer effectivement comme l'a dit la présidente Bruni de de garder une relation avec les territoires parce que lorsque bien une communauté de communes ou d'agglo créent des entreprises bien vous avoir une retombée et c'est tous leurs efforts, qui sera qui sera récompensé donc est-ce qu'il faut maintenir un CPE ou autre chose, mais je pense qu'il faut créer et conserver une relation avec les territoires, et peut être diminuée effectivement ou supprimé la la, alors en ce qui concerne la je pense qu'il ne faut pas effectivement augmenter les charges des entreprises, sinon, hé ben on aura des licenciements et des des des déficits et obligatoirement des, des, des licenciements dans les entreprises. Vous savez, tout à l'heure, on se demandait pourquoi nous n'avons, nous n'arrivions pas à affronter le problème du financement de la branche autonomie il y a exactement pour ce qu'on entend au jour en ce moment. Parce qu'au fond, vous ne le dites pas comme ça, mais pourquoi vous ne voulez pas financer véritablement. Une branche autonomie parce que ça coûterait beaucoup d'argent comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Pierre Sueur et ce beaucoup d'argent, il faudra le prendre sur les richesses créées par le travail, il n'y aura pas d'autre solution si nous voulons affronter ce problème de société qui est le problème de l'autonomie, il faudra aller chercher de l'argent, créée par le travail, si vous continuez à chaque fois qu'il y a un besoin devant nous un besoin de cette importance de dire ah oui, mais les charges des entreprises, on ne peut pas, parce que de quoi on parle quand on parle des charges, on parle des cotisations sociales, de ceux qui financent la protection sociale et qui fait que notre pays est est un pays compétitif. Un pays en bonne santé, parce que, heureusement qu'on met beaucoup d'argent dans la protection sociale ont heureusement qu'on met beaucoup d'argent dans la protection sociale, parce que c'est pour ça que ne les travailleurs de notre pays sont encore, encore aujourd'hui, et malgré tout, les dégâts faits. En bonne santé qu'ils peuvent encore prendre des retraites, et cetera, donc ça n'est pas une charge pour la société, c'est ça le progrès de la société et c'est parce que vous refusez de le financer, à la hauteur de ce qu'il faudrait que nous n'arriverons pas par exemple à financer la branche autonomie ou que nous créons des trous sans cesse dans le niveau de protection sociale des Français, notamment dans leur protection maladie pour les gens les plus défavorisés donc réfléchissez à ça parce que si à chaque fois que nous abordons ça le naturel revient au galop et que vous nous ressortez le discours sur ah la la, mais il y a beaucoup trop de cotisations sociales en France, hé bien les progrès de société, c'est-à-dire que nous devons faire, nous ne les verront jamais.

des emplois, des seniors dans l'emploi et de l'employabilité des seniors, c'est un amendement qui tient à coeur, pour Jean Marie Berg, donc il le proposer de créer un index senior pour observer la politique mise en oeuvre par les entreprises concernant l'intégration et le maintien dans l'emploi des seniors ainsi en deçà d'un certain seuil, qui sera défini en par décret en Conseil d'État, l'entreprise verra diminuer le bénéfice des exonération globale, battu de 10 pour % par ailleurs sans amélioration de cet index sur 3 ans, le montant total de l'exonération sera annulé au delà d'un certain seuil défini par le même décret l'absence d'évolution positive de l'index ne justifiera pas l'annulation de l'exonération je vous remercie. Oui merci, cher collègue, on sait que le travail de Jean Marie va leur Edberg sur ce sujet a été important, il le reste, c'est une de ses préoccupations et c'est forcément une préoccupation que nous par. Le maintien des seniors dans l'emploi, l'employabilité des seniors, ce sont autant de sujets sur lesquels la France n'est pas performante, il faut le regarder très honnêtement au niveau européen c'est c'est catastrophique je, je pense que les choses vont probablement changé parce que, aujourd'hui, il y a un manque de de d'offres et et je pense que toutes les entreprises recherchent de de la main d'oeuvre recherche finalement de l'expertise et l'expertise, elle se trouve aussi chez les seniors et j'espère que, en fait, ils en profiteront, il y a aussi le fait d'avoir augmenté le niveau de l'apprentissage dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de lieux et je pense que les anciens de l'entreprise ou de n'importe quel secteur d'activité ont des choses à transmettre et c'est important qu'on puisse y penser aussi, mais en tout cas le l'objet de cet amendement, je pense que nous y reviendrons quand tu nous parlerons avec René-Paul Savary de la proposition sur la réforme des retraites parce que dans finalement la la convention qui est proposé, la convention nationale, c'est l'une des pistes que l'on en fait en terme de réflexion aux partenaires sociaux et je pense qu'il faudra revenir à ce moment-là, et si c'est pas à ce moment-là, ce sera dans la future réforme des retraites que que vous proposerez probablement je je crois qu'il il est important de de revoir cet index comment finalement le construire et pour qu'il soit et et finalement opérationnel, donc c'est un avis défavorable pour l'instant, mais en fait, l'idée est excellente, merci. Merci, monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président sera une demande de de retrait sur cet amendement, puisque effectivement 2 occasions à venir pour pour discuter de ce sujet fondamental d'une part, comme l'a dit, la rapporteure générale les discussions autour de la réforme des retraites, d'autre part, puisque je comprends que que l'amendement s'appuie sur le dispositif ZRR la discussion que nous allons avoir sur la la génération suivante des ZRR dont le dispositif va venir en principe en en extinction et donc pour la question de son renouvellement de sa réforme à se poser pour cela, nous pourrons notamment nous appuyer sur le le rapport de de votre collègue Bernard Delcros, auquel j'ai pu contribuer

au moment où on va discuter de la réforme des retraites, l'employé militer des des seniors est une question absolument fondamentale parce que si on prolonge la durée de travail, c'est Jean-Marie vers le Rhône qu'il dure et qui le dit souvent et qu'en même temps, les seniors ne restent pas plus longtemps dans l'emploi dans les entreprises, évidemment il va y avoir un transfert sur la protection protection sociale et un transfert sur l'assurance chômage et puis un transfert sur le RSA et et puis un appauvrissement des, des, des, 10 senior et donc c'est une question fondamentale, mais on a bien noté que c'était pris en compte par la rapporteure générale et et par le ministre, je vous remercie. Merci monsieur le président, donc, cet amendement de nos collègues centristes reprend le dispositif d'un amendement déposé par notre groupe depuis des années, visant à réduire les les exonérations de cotisations sociales des entreprises qui ne signe pas d'accord relatif à l'égalité professionnelle ici l'amendement crée un index, emploi des seniors, des entreprises et réduit le montant de l'exonération en fonction du nombre de salariés en fait carrière, nous partageons l'idée que moduler le taux de cotisations sociales des entreprises peut avoir un effet un effet incitatif sur le comportement des employeurs et le maintien dans les effectifs des seniors, pour rappel, en 15 ans le taux d'emploi des seniors est passé de 38 à 56 % et demeure en dessous de la moyenne européenne, il faut inciter les employeurs à conserver les seniors dans les entreprises, plutôt que de les licencier à 55 ans, pour ces raisons, nous nous soutiendrons cet amendement et nous attendons le soutien de nos collègues centristes à notre amendement 769 examiner dans quelques minutes pour les entreprises ne qui ne conclut pas d'accord relatif à l'égalité professionnelle, je vous remercie. Très rapidement, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas traiter ce soir, l'emploi des seniors mais c'est véritablement ce qui fera réussir ou pas une future et pommes des retraites, je vois pas bien le rapport entre l'index et les ZRR,

ou qu'ils maintiennent pas l'emploi des seniors au sein de leur entreprise, il y a certaines sanctions qui peut être fait, mais je pense que le discours est prématurée, moi, moi je ne suis pas favorable à ce type d'un ex-parce que il faut définir déjà quel âge vous êtes le senior, après faudra pour l'embauche des jeunes Index, parce que si on embauche des seniors, on a, d'un point du des jeunes, donc c'est prématuré, attendons, nous attendons vos propositions sur l'emploi des seniors, c'est plus important, c'est un vrai sujet de société, faut changer l'oeil, la vision de la société sur les seniors, en conséquence, je pense que cet amendement est un peu prématuré simplement Jean-Marie Vollant 2 Arenberg souhaiter que on vous sensibilise sur l'emploi des seniors, ce qui est, au moins, chose faite, même si on ne vende pas, si on ne vote Oui merci monsieur le président, moi je ne rentrerai pas dans le dans le détail de cet amendement, mais je trouve qu'il a effectivement le mérite de, de, de placer cette question au centre du débat, vous nous répondez, Monsieur le Ministre, que la question, il sera étudiée voir régler lors d'un prochain projet de loi sur la réforme des retraites, moi je vais vous dire ce que je pense, hein, je pense que c'est une carotte. Qui nous est proposé pour nous faire valider cette idée de réforme des retraites et des carottes il y y en aura d'autres, on va nous parler des carrières des femmes, enfin des retraites des femmes : on va nous parler de l'emploi des seniors, on va nous parler de 2 ou 3 autres sujets comme ça des, des, de la pénibilité qui a été dont les critères ont été supprimés, il y a tout juste 2 ou 3 ans sous le mandat précédent, l'emploi des seniors, on ne le résoudra qu'avec les entreprises, le risque durera pas à coup de textes votés ici on le résoudra par des contraintes certainement alors pas que des contraintes, mais il faudra une partie de contraintes, on se rend compte ici que lorsque l'on veut mettre. évoquer certaines, certaines questions et notamment par exemple, trouver des solutions financières pour la branche autonomie ou comme ça, ça passe par des contraintes aux entreprises, c'est-à-dire des cotisations supplémentaires et c'est toujours non c'est toujours non c'est toujours non, moi, vous savez sur cette histoire d'emploi des seniors, je ne crois que ce que je vois, mais je vous avoue que j'ai énormément de doutes. Collègue, Monsieur le Ministre, vous souhaitiez apporter quelques précisions. Des retraites. Monsieur le président, vous vous êtes sûr parce que je, je m'apprêtais à me lancer dans une

ou d'exonération plutôt qui concerne les zones de revitalisation rurale c'est peut être pas l'intention de l'auteur, mais c'est ce qui est écrit. Merci, Monsieur le Ministre, donc je mets aux voix l'amendement 144 avec 2 avis défavorable qui est pour.

Merci monsieur le président, alors le GIEC comme l'ONU comme les ONG environnementales sont unanimes : il est plus que jamais urgent de limiter les effets de nos sociétés sur le climat sur la planète pour cela plusieurs façons de procéder, en termes de politique coexistent, qu'il s'agisse de contraindre ou d'inciter, il faut vite tourner la page du système productiviste dans lequel nous vivons au profit d'une société respectueuse de l'environnement et des limites fini de la planète, c'est pourquoi cet amendement vise, dans une logique incitative à conditionner pour les multinationales, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de contreparties écologique indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique, les enjeux en la matière, sentiment s'sont connus en mars 2021, l'ONG Oxfam Oxfam révélait que les activités industrielles des multinationales nous parlons dans cet amendement, c'est les multinationales du CAC 40 nous conduisent vers vers un réchauffement planétaire de plus 3 virgule 5 pour ce degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ces entreprises doivent impérativement participer à la transition et réduire leur émission de gaz à effet de serre pour leur prise de conscience rapide désormais et afin de les inciter à participer à la lutte contre le changement climatique, nous proposons de conditionner les avantages sociaux dont elle bénéficie, est largement actuellement alors prise en compte des indicateurs environnementaux, quand je dis nous, c'est bien sûr les écologistes mais de plus en plus ce sont des institutions internationales et nationales qui exige la conditionnalité des aides, des subventions aux entreprises, à l'engagement, notamment d'être dans la trajectoire de l'accord de Paris merci. Oui, alors nous, c'était un amendement qui a, qui est dans le même esprit, nous proposons pour les les très grandes entreprises, les exonère que les exonérations de cotisations patronales à l'assurance maladie soit conditionnée à trois critères cumulatifs vertueux la fixation d'une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, l'absence de délocalisation à l'étranger et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Merci, cher collègue, le 718 Madame Poncet Monge. merci Monsieur le Président, ben, cet amendement, de nouveau, a pour objet de conditionner pour les multinationales, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de contreparties écologique et sociale en 2020 la transformation du CICE on a le on allégement pérenne de cotisations patronales a représenté un coût de 22 milliards d'euros pour la sécurité sociale, compensé par le budget de l'État, à l'époque on parlait d'un million, il y avait un pinceau d'un 1000000 de créations d'emplois, effectivement, vous nous avez dit un million, mais ça a pas été en 2 lors de la création, c'est donc une dépense publique en plus de son coût exorbitant, il a été établi que cette politique était inefficace en matière de création d'emplois, je crois qu'elle a créé 350000 emplois, je vous laisse faire la division du coup de chaque emploi aussi au regard du coût financier de ce dispositif à l'utilité économique très contestable et contestées par les par les organismes de statistiques, nous proposons un dispositif cumulatif permettant de s'assurer que ces allégements présente une réelle utilité pour notre société, en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, l'enjeu est immense, loin des engagements des accords de Paris la trajectoire actuelle, il est bon de le redire de température, conclut à une hausse globale compris entre et cinq 7 en 2050 selon le GIEC, une planète à 5 degrés être tout simplement inhabitables pour l'humanité, très récemment, le secrétaire général de l'ONU, alertait en le 28 octobre dernier le monde file vers une catastrophe mondiale, tout en s'indignant les engagements des États ne sont pitoyablement pas à la hauteur, ainsi, c'est parce que notre société se trouve actuellement au coeur de défis socio-écologiques critique que nous devons enfin adopter des mesures incitatives afin d'accélérer la mise en oeuvre des transformations nécessaires pour l'instant par l'ensemble des acteurs de la société. Le 722 s'il vous plaît, si vous pouvez enchaîner avec le 722. Nouvelles il est bien défendu. Allez défendu merci madame pour ce monde. Madame la rapporteure. merci Monsieur le Président, chers collègues, en fait, à travers tous ces amendements, vous proposez de conditionner en fait les allégements généraux au respect de diverses qu'en contrepartie climatique et sociale et sur les 2 premiers amendements qui sont les mêmes d'ailleurs, je voudrais simplement vous dire que c'est assez Important en termes de conditions là c'est pas une condition mais c'est plusieurs que vous mettez dans cet amendement et ça instaurerait je pense pour les entreprises des contraintes et des contrôles très très lourd et sans doute une une forte insécurité juridique, c'est donc un avis défavorable sur les 2 premiers pour le suivant de Madame Poncet mange le numéro 723 les obligations qui sera TiVo au climat ne relève pas de la politique de la sécurité sociale, les incitations et les sanctions relatives à ce domaine gagnerait à être abordée dans un autre cadre, c'est donc aussi un avis défavorable sur l'amendement qui n'a pas été forcément exposé, je vais être un petit peu plus longue, les entreprises disposant d'une ou plusieurs sections syndicales ont l'obligation d'engager tous les 4 ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est déjà une condition d'ailleurs dans l'amendement de Madame Lubin, à défaut d'accord, l'employeur doit établir un plan d'action annuelle destinée à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une sanction, vous le savez, pour la plupart déjà prévues pour les entreprises d'au moins 50 salariés qui ne respectent pas ces obligations, elle s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de leur masse salariale, si elles n'ont pas régularisé leur situation, un mois après la mise en demeure de l'inspection du travail qui a constaté le manquement en pratique, les services du ministère du Travail m'ont indiqué que dans une très large majorité des cas, les mises en demeure sont suivies d'une régularisation de la situation et qu'elle ne donne pas lieu à pénalité en 2020 35 pénalités ont été prononcées sur 198 mise en demeure, les entreprises tendent donc à régulariser leur situation après le contrôle de l'inspection du travail, ce qui montre que le dispositif est déjà incitatif depuis l'entrée en vigueur du dispositif de pénalités en 2010 et jusqu'à janvier 2021 358 pénalités ont été prononcées pour un montant moyen de 14000 euros par pénalité c'est pas rien, le dispositif semble donc efficace et respecté, ce qui laisse penser que les sanctions déjà prévues s'avère suffisante pour inciter les entreprises à négocier sur l'égalité professionnelle, bien que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes demeurent significatifs, les sanctions des sanctions supplémentaires ne semble donc pas ce que vous proposez n'est pas le levier le plus pertinent pour assurer l'égalité des rémunérations dans les entreprises, c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Bonjour, monsieur le président, oui, merci, moi je voulais venir en soutien cet amendement parce que on a eu au début de la discussion un amendement qui était similaire qui visait aussi à imposer une conditionnalité des aides aux entreprises qu'on été environnementale, sociale on nous a dit que c'était trop flou assez opérationnel, là on a un amendement qui est très opérationnel, il concerne les très grandes entreprises, c'est environ 250 entreprises en France qui touche environ un tiers des, des, des, des exonérations de charges dont on parle, et des critères très précis, alors vous êtes peut-être pas d'accord, mais ils sont quand même très précis, très opérationnel, et moi je trouve que quand on a tellement d'appétence à aller contrôler les millions de personnes qui touche 598 euros par mois pour savoir qu'elle les dépense bien quand on a autant d'appétence allait contrôler que celles et ceux qui touchent l'allocation de rentrée vont bien dépensé pour les gommes et les crayons et pas pour les tablettes et quand on a autant d'appétence allait contrôler que les associations dépense bien en subventions comme il faut et qu'elles font bien les audits qu'il faut, là on a 250 entreprises qui touchent des milliards et dont on doit juste savoir est-ce que la solidarité nationale profite à des entreprises qui ont des activités qui nous mettent sur le chemin d'un monde vivable, ou sur le chemin d'un monde invivable et on dirait : ah ben non, on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir si les dizaines de milliards qu'on dépense, ça sert à ce que le monde soit vivable ou invivable à ce que le monde soit juste ou injuste, moi je, je comprends pas, je trouve que c'est, c'est c'est de la mauvaise gestion.

en tout cas, il y a un autre amendement de repli, alors là, on ne va pas parler du du du mode de de ma vivable, on va juste parler de quelque chose qui encore et et encore plus parlant pour vous, immédiatement, c'est en fait de conditionner le bénéfice des allégements au respect de l'absence de délocalisation et de l'égalité salariale entre femmes et hommes, le fait de ne pas délocaliser et le fait de tendre à l'égalité salariale entre femmes et hommes et partager ici sur ces bancs, par tout le mode la rapporteure, nous a dit, pour l'égalité, ce n'est peut-être pas le meilleur levier certes, cela étant dit, voilà la rapporteure je bascule de vous dire qu'il peut y avoir plusieurs leviers, il y a des leviers qui fonctionne, il fonctionne pas encore suffisamment puisque les femmes gagnent encore en moyenne 22 % de moins que les hommes donc actionnant d'autres leviers avec lesquels vous êtes fondamentalement d'accord sur le résultat que nous devons obtenir et qui ne touche toujours que le même nombre d'entreprises que ce que vient d'expliquer Mélanie Vogel. Donc ça c'est le le 722. c'est juste pour attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que si justement on conditionnait les aides publiques. Que l'on accorde aux entreprises, il y aurait un gain pour notre économie, pour notre service public, et cetera de 100 à 200 milliards d'euros, alors je pense que les amendements de nos collègues d'Europe Écologie-les Verts qui ont en fait cette orientation serait très positif pour toutes et tous. Merci, cher collègue, donc je mets aux voix le 721 avec 2 avis défavorables est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le pour le 1048 avec 2 avis défavorables même vote même vote il n'est pas adopté même vote pour 723 même vote il n'est pas adopté même vote pour 722 il n'est pas adopté, nous passons à 2 amendements identiques, le 700 pardon il est un peu plus de minuit, je vous propose de prolonger jusqu'à une heure du matin notre séance

Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plus de 20 ans, les exonérations des cotisations sociales accordées aux entreprises connaissent une croissance rapide, sobre, sans transparence et ni conditionnalité, selon le dernier rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, publié en 2022, la participation des employeurs privés au financement de la Sécurité sociale est devenue minoritaire alors qu'en 1990 leur part été de 51 %, celle-ci est tombée à 36 de 5 pour 100 en 2019 ainsi l'effort contributif des entreprises n'a cessé de se réduire, tandis que les prélèvements sur les ménages n'ont cessé de croître, il en est ainsi de l'allégement de cotisations patronales d'assurance maladie, qui représente un coût annuel moyen de 22 milliards d'euros pour l'assurance maladie, sans contrepartie, et dont l'efficacité en termes de création d'emplois est loin d'être démontré, nous proposons donc de poser des conditions à l'allégement des cotisations patronales, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'interdiction de délocaliser des activités à l'étranger si cela entraîne une diminution du nombre d'emplois en France et la remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, merci. Oui, les amendements que vous proposez, revient à une subordination, une nouvelle fois des conditions de la réduction de cotisations maladie jusqu'à 2 5 du SMIC au respect de diverses conditions sociales mais cette réduction en fait de cotisations maladie à remplacer le CICE je pense que vous le savez, mesures de compétitivité qui n'était pas subordonnée à de telles conditions, donc c'est un avis défavorable de la commission. Merci, monsieur le Ministre, même avis ma vie. Donc je mais on voit ces deux amendements identiques le 1679 et 1049 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés le 1047 Monsieur Jomier. Merci monsieur le Président, la question des exonérations pose la question de leur pertinence et leur efficacité, le Conseil d'analyse économique, dans une note publiée en 2019 confirmé d'abord que les baisses de cotisations sur les bas salaires inférieurs à 1 1 1 virgule 6 fois le SMIC, produisent des effets au soutien de l'emploi et de la compétitivité des entreprises, mais recommandé également l'abandon des exonérations de cotisations sur les salaires supérieurs à 2 5 fois le SMIC au motif motif qu'elles sont sans effet sur l'emploi et la compétitivité principalement sans incidence sur les exportations de ces entreprises et à l'inciter les pouvoirs publics à remobiliser ses fonds sur des la suppression des impôts, de production tout cet amendement pour exactement sur une de ses Oeuvres exonération en proposant la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales pour les rémunérations comprise entre 2 virgule 5 et 3,5 fois le SMIC et à travers cet amendement, nous voulons donc que s'ouvrent le débat sur l'adaptation des exonérations à leur efficacité après une évaluation. Je je je veux notamment relevé que cet amendement a été déposé à l'Assemblée nationale, par 25 députés du groupe Renaissance, dont le président de la commission des lois dont la porte-parole du groupe Renaissance et que le gouvernement n'ayant pas été content de ce dépôt, probablement, il a été retiré mais ça veut bien dire que le débat doit être ouvert et que ce débat, le Parlement doit s'en saisir ces 71 milliards d'exonérations ne sont pas un ensemble homogène, certaines sont utiles, d'autres non, acceptons d'aller les évaluer et de supprimer celles qui n'ont pas d'intérêt pour l'emploi pour l'emploi et pour l'activité économique, c'est l'objet de cet amendement. Madame la rapporteure. Oui, il y a quelques minutes, nous étions sur les la réduction des cotisations maladie et et là on est sur les cotisations familiales, donc c'est une limitation de la réduction de cotisations familiales à 2 5 SMIC je pense que a minima, c'est vrai qu'il faut avoir le débat mais sans doute faudrait-il aussi avoir une étude d'impact sur les effets d'une telle mesure, même s'il y a une certaine logique, comme vous l'avez dit à réserver ces exonérations et ces réductions de cotisations à des salaires bas ou moyen, c'est, c'est c'est la réalité, vous le vous l'avez très bien n'exprimer mais la commission a un avis défavorable sur. Même avis pour Monsieur le Ministre Monsieur Jomier. Merci monsieur le président, mais brièvement le gouvernement n'apporte là, aucune réponse est-ce que vous êtes gêné est-ce que vous pouvez envisager au moins l'étude sérieuse de ce de la suppression de ce type d'exonération voir avec une progressivité, je veux dire on on peut comprendre, mais là on n'a aucun mot du ministre, alors que la proposition mérite d'être discuté, moi je le regrette vraiment.

sous la peine bah on va avoir des exonérations de côté de cotisations sur les bas salaires, donc ça fait baisser en même temps, le coût du travail, je vous le rappelle, quand même, mais en même temps de nombreuses heures supplémentaires sont mis en place et ça ne crée pas forcément de l'emploi, donc je pense qu'il faudrait vraiment, regardez, il faut que, qu'on prenne conscience de l'impact, si réellement ces examens ces exonérations valent le coup au niveau de la population française, merci.

oui, je trouve que la réflexion de notre collègue Bernard Jomier et tout à fait acceptable et d'ailleurs je, je vois que dans son amendement, il confirme bien que les baisses de cotisations ont été importantes, produit des effets au soutien de l'emploi et de la compétitivité des entreprises, bon, je pense que ça c'est déjà très bien et, par contre, je pense que y'pourquoi ne pas avoir une réflexion pas un rapport mais au niveau de l'État pour savoir effectivement quels sont les réductions de charges enfin de cotisations, excusez-moi, j'ai dit charges c'est vrai faut des réductions de cotisations qui rende pleinement ce que nous cherchons, c'est-à-dire, création d'emplois pour qu'il y ait davantage d'employer davantage de cotisations pour notre système social. Merci, merci, cher collègue Madame pour ce monde. Très rapidement, on dirait qu'il y a pas eu de d'étude de l'Insee sur par exemple les emplois créés par le CICE, enfin je veux dire, elles existent, elles sont effectivement les effets sur l'emploi sont ridicules, ce que je crois que c'est 350000 emplois bien donc cela existe et moi ce que je voudrais remarquer c'est c'est que quand on baisse les cotisations, quand on demande des exonérations tout azimut, là il y a pas d'étude d'impact, hein, bon et puis quand on dit qu'on veut supprimer une partie assez quand de Bernard Jomier, hé bien là, on dit : il faudrait une étude d'impact, hein, quand on baisse quand on fait des exonérations, pas besoin d'étude d'impact quand les évaluations Insee sont là, et bien on n'en tient pas compte, mais par contre qu'on veut remettre en cause ces exonérations nous dire bon connaît pas bien l'impact non c'est quand même enfin. C'est un Merci monsieur le Président, simplement rappeler que ce cette exonération ce bandeau familles ces 2015 et c'est le le le gouvernement de François Hollande qui l'a qui l'a institué, bon, on a le droit de se tromper, c'est la raison pour laquelle il est important qu'il puisse y avoir des évaluations de chacun de nos dispositifs des niches fiscales et des niches sociales. Dans la nouvelle loi organique de financement de la Sécurité sociale, il y a désormais un rythme de tous les 3 ans auxquels les niches sociales sont sont évalués et donc c'est c'est au printemps prochain, au printemps 2023 que sera le le le rapport triennal de d'évaluation des niches sociales ce qu'à l'occasion d'avoir ce ce débat sur l'efficacité, en l'occurrence du du bandeau famille. Merci, monsieur le Ministre je mais aux voix l'amendement 1047 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Attendez, on va faire un debout, assis, je suis désolé, qui est pour se lève. Merci qui est contre, se lève. merci qui s'abstient se lève. Donc il n'est pas adopté cet amendement discussion commune dans 2 identique le 724 madame Poncet mange. C'est monsieur le président, la crise sanitaire que nous traversons, donc depuis 2020, a eu pour conséquence une forte dégradation du solde de la Sécurité sociale, le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, bon je passe les chiffres mais les prévisions pour les années suivantes sont très incertaines puisqu'elles dépendent aussi de l'évolution de la situation sanitaire et de l'économie mondiale en matière d'accès aux soins, la politique d'investissement doit se poursuivent pour combler le sous-investissement depuis plus de 20 ans diminuer sensiblement le taux de vétusté, je parle notamment de l'hôpital public, renforcer la résilience de système de santé face au changement climatique oh possible pandémie, nous sommes entrés dans l'ère des pandémies et préparer l'ensemble du système de soins affronter le changement démographique depuis 2013 jusqu'à sa suppression en 2019 le CICE représenter une perte de recettes annuelles de près de 22 milliards d'euros, je l'ai déjà dit pour les pour les comptes de l'État, avec une certaine inefficience de ce dispositif, pourtant été transformée depuis en une réduction des cotisations patronales, qui représente un manque à gagner important pour les recettes de la Sécurité sociale qui sont pas toujours compenser totalement cet amendement vise donc à abroger les dispositions introduites par l'article 8 de la loi 2018 12 103 du 22 décembre 2018 et concrétiser au sein du code de la sécurité sociale à travers l'article L 241 13. Merci amendements identiques le 1668 Madame Cohen. Oui, monsieur le président, les allégements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires représentent en 2021 83 % du montant de l'ensemble des mesures d'exonération de cotisations et contributions de Sécurité sociale, ils comprennent 3 dispositifs juridiques distinctes, la réduction générale dégressif jusqu'à 6 SMIC applicable depuis 2005 qui permet d'exonérer au niveau du SMIC, la totalité des cotisations et contributions obligatoires, la réduction de 1 virgule 8 points des cotisations d'allocations familiales sur toutes les rémunérations inférieures à 1 virgule 6000 en 2015 et 3 5 SMIC depuis 2016 versée par les employeurs éligibles à la réduction générale dégressive, la réduction de 6 points des cotisations d'assurance-maladie, sur toutes les rémunérations inférieures à 2 5 SMIC versée par les employeurs éligibles à la réduction générale dégressive

soit plus que les suppressions de cotisations du CICE qui coûte 24 5 milliards d'euros, quel gâchis, quel argent perdu, qui ne peut que faire défaut aux hôpitaux, secteur de la santé au secteur médico-social et ces exonérations qui grèvent le budget de la Sécurité sociale et ampute également le budget de l'État qu'il les compense en partie, on peut se demander quel effet elle et et ils ont les rapports sont unanimes pour dénoncer ces exonérations qui contribue à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification alors, mes chers collègues, Stop ou encore les exonérations.

elle est conditionnée à des pratiques en matière d'emploi, de salaires, d'investissement ou d'impact sur l'environnement pratiques vertueuses bon, toujours le même type d'amendements. Chers collègues, le 769 Madame Cohen. Oui, le fossé entre le salaire horaire brut moyen des femmes et des hommes ne serait job que font lentement malgré les lois successives en matière d'égalité professionnelle, selon une étude du ministère du Travail, réalisée auprès de 40000 entreprises françaises de plus de 50 salariés, seuls 6 % d'entre elles versent des salaires égaux pour leurs employées pour les entreprises de 1000 salariés, seul 1 % d'entre elles sont exemplaires, il nous semble important d'aller plus loin que les mesures qui t'ont qui ont été prises contre les inégalités salariales, nous sommes en 2022, mes chers collègues, il est grand temps que l'égalité progresse progresse et que la République soit à la hauteur de son principe d'égalité, il faut au minimum conditionner les aides aux entreprises à des critères d'égalité stricte et encadrée, une différence entre les entreprises vertueuses, il en existe quelques-unes et celles qui ne respectent pas la loi est absolument nécessaire, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une telle situation inégalitaire entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, ainsi, à partir du 4 novembre à neuf heures 10, les Françaises travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, je pense que nous serons d'accord pour nous dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire de la loi telle qu'elle est actuellement écrite il faut opter pour une autre approche afin de garantir une égalité salariale effet. Steve entre les hommes et les femmes avec cet amendement, c'est ce que nous proposons la responsabilisation par la pénalité nécessaire, nous vous rappelons que l'égalité entre les hommes et les femmes est érigée en priorité interministérielle, soyons donc dans l'action et la responsabilité mais aussi et surtout soyons cohérents, d'où la nécessité de voter notre amendement. monsieur le président, mes chers collègues, donc cet amendement prévoit qu'en France les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes, on estimait à 2017 qu'à partir du 3 novembre. En raison des inégalités salariales, les femmes travailler bénévolement jusqu'à fin l'année elles représentent 80 % des travailleurs pauvres et à la course après que la précarisation, les touches de points plein fouet malgré les lois successives en matière d'égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire c'est ce de se réduire à ce constat, cet amendement propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leur obligation en matière d'égalité salariale. Oui, merci Monsieur le Président, alors ça a été dit le le fameux jour où les femmes effectivement cesse d'être payé comme les hommes, c'était le 3 novembre à neuf heures 22 pour être précis, le jour de dépassement de des limites écologiques qui, chaque année, plus tôt, c'était le 28 juillet maintenant, nous avons 2 jours de dépassement par année. Le jour de dépassement écologique 28 juillet le 3 novembre le jour de dépassement de l'égalité femme alors vraiment l'égalité salariale quand même, et non seulement nécessaire, par principe, hein, nous serons d'accord mais elle améliorerait en plus les conditions de vie, de nombreuses personnes et permettrait aussi de renflouer les caisses de Sécurité sociale si les femmes étaient payées comme les hommes, alors moi je sais pas, c'est un chiffre que j'avais, que je n'ai plus mais je crois que là, le déficit de la Sécurité sociale, ça serait terminé, hein, et donc la mesure que nous proposons, elle est dissuasif pour les entreprises non ça ne va pas assez vite, madame la rapporteure générale, je suis désolé et et il est temps, vraiment, de permettre de progresser beaucoup plus vite, c'est un peu comme l'écologie dans la juste lutte contre les inégalités femmes-hommes et contre la culture patriarcale, il faut bien le dire, pour nommer les choses. la suppression pure et simple des allégements généraux ça aurait pour conséquence, 25 milliards d'euros sur le coût du travail supplémentaire, donc c'est énorme à un moment où justement les entreprises affronte des difficultés de par les frais d'énergie le frais de, les frais de matériaux, etc donc je pense que c'est c'est pas le bon moment de, de, de proposer, hein, une telle suppression pour les autres qui sont sur la condition de l'égalité homme-femme, je crois, Me exprimé en détail tout à l'heure. Monsieur le Ministre, même avis. Donc je mais aux voix les amendements 724 et 1668 identique monsieur Milon oui très court, s'il vous plaît parce que faut qu'on avance là quand même monsieur, monsieur le président, mais je vais essayer d'être court mais j'ai, j'ai 2 minutes, donc ça va, ça fait 120 secondes non, je voulais juste rappeler certaines choses qui ont été dites dans le cas de de de ces amendements particulier par par rapport à ce qu'a dit Raymond pose mon nous ne sommes pas c'est dans ce siècle rentrer plus dans le monde de la pandémie que dans les siècles précédents, certes, on a eu la Covid et on a maintenant les bronchiolites, mais dans les siècles précédents, il y a eu la grippe espagnole a eu la grippe et sciatique, il a eu la diphtérie et dans les siècles qui était passé dans il y a eu la peste, et

Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés je mets aux voix le ML avec 2 avis défavorables qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 769 2 avis défavorables même vote même vote il n'est pas adopté le 1033 même vote il n'est pas adopté. Le 162 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 718 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 765 Madame Cohen. Dans le monde scolaire. Madame pour ce policier. Merci monsieur le président, mes chers collègues, je vais vous proposer ici un amendement qui va certainement être voté majoritairement voire unanimement puisqu'il s'agit des grandes entreprises françaises qui ont versé au cours du 2ème trimestre 2022 des dividendes à des niveaux encore jamais atteint, faut-il le rappeler, 44 3 milliards d'euros, soit 33 % de plus par rapport à 2021 en France, je rappelle que ces entreprises du CAC 40 ont bénéficié pendant la pandémie de près de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État de 110 milliards d'euros dans le dans le cadre du plan d'urgence de baisses d'impôts, d'une aide de 100 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance du chômage partiel pour 31 milliards d'euros, des reports ou annulations de cotisations et de charges fiscales pour 76 milliards d'euros et des les entreprises en persillade de crise se justifie quand il s'agit des plus fragiles, mais pas celle du CAC 40 qui profitent de la crise pour réaliser évidemment encore plus de bénéfices dans la mesure où ces entreprises ont bénéficié du filet de sécurité de notre sécurité sociale, il serait parfaitement logique de soumettre à cotisation sociale, leurs revenus financiers face à un contexte inflationniste et de crise énergétique inédit mais également face à la nécessité, trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires au taux actuel des cotisations sociales employeurs de la sécurité sociale, il s'agit aussi d'une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail je vous remercie. Oui, je pense que notre collègue était optimiste, elle sait que la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cette proposition, une proposition qui concerne en fait toutes les entreprises, et pas seulement celles qui font comme on ne l'a dit hier des super profits donc malheureusement c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre.

de petites PME pour lesquelles le dividende est une modalité une modalité principale de rémunération et puis y a les 3 millions de salariés actionnaires qui qui se verrait frapper pour les les distributions d'une d'une d'un taux de prélèvement de 70 %. Merci donc je mets aux voix le 765 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 3 amendements identiques, le 725 Me Poncet Monge. Merci monsieur le président, c'est à cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations sociales ou des socialisation de des heures supplémentaires, en vigueur depuis 2019, cette mesure a été renforcée par les mesures d'urgence économique et sociale, elle est souvent souvent présenté à tort comme une mesure de partage de la valeur pour les Français depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires sont exonérés de cotisations sociales salariales, dans la limite d'un taux de 11,31 % d'impôt sur le revenu, jusqu'à un certain plafond, depuis la loi de finances rectificative pour 2022, celle-ci a modifié le seuil d'exonération fiscale qui est désormais fixé à 7500 euros à plusieurs égards, ces exonérations pose problème au, delà de représenter un manque à gagner et pour les finances publiques des incite au recrutement en encourageant les employeurs à s'appuyer sur les heures de travail supplémentaires de leurs employés en poste ensuite ces exonérations représentent une baisse du prix du travail et de la rémunération brute des salariés, enfin et surtout, je dirais, en encourageant ces mêmes salariés effectuer plus d'heures, ce souvent d'ailleurs pour simplement maintenir leur pouvoir d'achat érodé par l'inflation, elle pousse à l'épuisement professionnel et vont à l'encontre d'objectifs écologiques de baisser le temps de travail pour travailler mieux et tous oui, le droit à la paresse, avec 7500 d'heures supplémentaires, allons ainsi ce dispositif pousse les salariés à travailler davantage, ou les oblige les les oblige au détriment de la création dans. Quoi, mais surtout de la promotion de la santé au travail et de la prévention des risques psychosociaux.

Alors cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires, la mesure instaurée en 2019 consiste en une exonération de la totalité des cotisations salariales du sur les heures supplémentaires et complémentaires effectués rémunéré sont exonérés des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaires plus concrètement encore ce dispositif entraîne une perte de recettes de 1 milliard 9 par an pour la sécurité sociale, d'après le ministre de l'économie, dans une réponse faite à la question écrite d'un sénateur en mai 2021, il faudra un jour que ce gouvernement s'explique du mécanisme qui le pousse à croire que renforcer le pouvoir d'achat passe par saper la protection sociale dans son autonomie financière et ainsi limiter sa capacité à répondre aux besoins sociaux, on trouve dans la presse ces chiffres d'un cas de 50 euros par mois pour un salarié qui touche 1500 euros mensuels ou 13 euros pour un salarié au SMIC, on espère que ce salarié ne doit pas s'acquitter d'un forfait patient urgences le FPE, d'après l'ouvrage annuel de l'adresse, minima sociaux et prestations sociales, les prestations sociales ont diminué, le taux de pauvreté de 7 6 points en 2019 de la même manière le nom tant de nos concitoyens et concitoyennes qui renoncent aux soins et aux prestations sociales malgré un emploi devraient nous convaincre de ne jamais opposé le salaire immédiat, pouvoir d'achat et le salaire socialisé cette part mutualiser qui réalise l'ambition d'un seuil de bonheur social qui nous anime encore si ces idéaux, nous ne vous convainc pas mes chers collègues prenons la note de l'économiste Éric Heyer, directeur du département analyse et prévention de Sciences Po, qui notait que l'effet négatif : hausse du temps de travail et perte d'emploi d'une telle mesure sur l'emploi, l'emporterait légèrement sur l'effet positif gars du pouvoir d'achat et de compétitivité, merci. Merci le MLI madame. Alors c'est le même, donc je ne développerai pas les mêmes arguments, je dirais simplement en complément qu'il est difficilement compréhensible de de voir que, moment où nous nous interrogeons pour savoir comment nous allons financer un certain nombre de choses, notamment l'autonomie, enfin, on en a suffisamment parlé la branche autonomie chaque fois qu'un dispositif est en en matière de, de, d'heures supplémentaires, il est systématiquement c'est c'est c'est tout à fait incompréhensible et à certaines périodes et nos. Notamment la période que nous vivons de plein emploi, il est totalement incompréhensible que l'on incite des gens à faire des heures supplémentaires des défiscalisé, j'avoue que j'ai entendu un mot qui ne va pas plus le droit à la paresse, chers collègues, les gens qui font des heures supplémentaires sont rarement des paresseux. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Oui c'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements, en fait, cet Avantage, il avait été comment créer par instauré par la loi Tepa de 2007, il n'a pas été supprimés entre 2012 et 2017 je pense tout au contraire de vous qu'il apparaît encore plus pertinent de de maintenir cet Avantage en période de tension sur le marché du travail dans de nombreux secteurs. Voilà. Merci même avis pour Monsieur le Ministre, défavorable, donc je mais on voit les 725 789051 monsieur Bena Ross. Oui, juste une seconde, je, je, je voulais me réjouir déjà que nos collègues les citer le droit à la paresse, très beau livre de Lafarge, qui était le gendre de Karl Marx, vous le savez peut-être, bon et je voulais rajouter une chose la, la, la réduction du temps de travail ou la répartition du temps de travail tout au long de sa vie ou, tout au long d'une semaine de mois par travailleur, c'est pas de la paresse, c'est la possibilité de s'occuper d'autre chose que de travail salarié d'avoir d'autres activités comme nous en avons tous d'ailleurs, c'est la possibilité de s'occuper de sa famille, de s'occuper de culture, de s'occuper de bénévolat, de s'occuper de beaucoup de choses qui sont absolument le contraire de la paresse, mais qui sont le symbole d'une intégration dans une société solidaire. Qui est contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés, nous passons à l'article 11 bis, l'amendement mais 52 madame Dumas. plus favorable applicable aux entreprises de moins de 20 salariés, notre groupe s'oppose à une disposition qui aura pour résultat de réduire les cotisations versées à la Sécurité sociale sans compensation par ailleurs cet article vient modifier des dispositions adoptées à l'été 2022, ce qui contribue à une instabilité qui donne une politique de gribouille qui n'est favorable ni aux institutions, ni aux entreprises ni aux citoyens. Merci madame la rapporteure. L'avis est défavorable parce que en fait il est contraire à la position de la commission qui a soutenu la réduction de cotisations au titre des heures supplémentaires pour les entreprises de 20 à 249 salariés je voulais aussi rappeler que c'était notre collègue, Frédérique Puissat, qui avait en fait défendu ce dispositif lors d'une précédente loi merci. Le ministre-défavorable aussi. Je mets aux voix l'amendement 1000 sac pardon madame pour ces manches. Très rapidement par rapport à l'argument comme quoi il y a des tensions sur le marché du travail si j'entends bien, si je comprends bien cet argument, ça veut dire que on préférerait bien embaucher des gens plutôt que de faire faire des heures supplémentaires, mais on ne trouve pas de personne, et cetera, et cetera, hé bien, si on devait embaucher des gens on paierait des cotisations salariales et patronales, je dirais même que, en période de tension de du marché de l'emploi si les heures supplémentaires sont substitutif de création d'emplois, faute de salariés enfin foutre d'offreurs de travail, hé bien, c'est un argument vraiment supplémentaire pour dire qu'il y a aucune raison, enfin c'est pas de c'est totalement de l'opportunisme, je parle de de l'exonération est pas de la rapporteuse générale de dans ce cas-là, d'exonérer de cotisations salariales et patronales. Merci donc je vais au voit le 1052 et 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté le 44 de la commission madame la rapporteure. Oui, alors, comme je le disais, je propose un amendement sur la réduction de cotisations sociales au titre du rachat de RTT effectués par les mêmes salariés avant le 31 décembre 2025, en fait, ce qu'on a accordé au titre de la réduction des cotisations sociales. Pour les heures supplémentaires, en fait, on va jusqu'au bout du processus et on prend aussi les RTT, en effet, je pense qu'il est illogique que pour ses seules entreprises le traitement fiscal et social des heures supplémentaires et des achats de RTT ne soient pas identiques, il est d'ailleurs probable qu'il s'agisse d'un oubli en fait les textes ayant institué ces 2 dispositifs ayant été en avaient en même temps, de plus, cet amendement codifie l'article 2 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ce dispositif présentant un caractère pérenne. Merci, monsieur le Ministre. ou le régime d'exonération a été étendue des entreprises de 20 à à à 250 salariés pour les heures supplémentaires et le principe de la monétisation. Des RTT a été acté. des, des groupes de groupes parlementaires de de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce que vous proposez c'est d'exonérer la part patronale de la monétisation des RTT, ce qui nous, nous paraît pas poursuivent l'objectif qui était poursuivi par l'idée initiale qui était de rang du pouvoir d'achat aux salariés. La la la la la la. L'exonération de la part patronale n'a pas de raison de de rende du pouvoir d'achat aux salariés, c'est la raison pour laquelle la position du du gouvernement et est défavorable sur cet amendement.

comment dire amélioration de pouvoir d'achat, c'était extraordinaire, donc effectivement il ne manque plus, pour couronner le tout, que d'exonérer tout cela de charges sociales patronales, salariales défiscalisation tout ça et tout va très bien. Merci, cher collègue dont je mais aux voix l'amendement de la commission de 44 avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre.

Merci monsieur le président, donc nous proposons par cet amendement, de créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant 5 plafond annuel de la Sécurité sociale vous pouvez faire le calcul afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale, enfin un rappel historique, en mars 1944 le Conseil national de la Résistance propose dans son programme, bien écoutez le CNR on en plat, de façon indue, donc ça me permet de de redire qu'il a un vrai CNR qui s'appelait le Conseil national de la Résistance. Qui propose dans son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer, pas de travail, les ordonnances des 4 octobre et 19 octobre 1945 créer une organisation de la sécurité sociale qui garantit à chacune et à chacun disposer en toutes circonstances, des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance, ainsi que celle de sa famille, dans des conditions décentes, selon un rapport, Oxfam, les 5 premières fortunes de France, les 5 premières ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie, elle possède à elle seule autant que les 40 les plus pauvres de France, les quatre premiers décide, c'est bien que si il serait possible de quadrupler quadruplé le budget de l'hôpital public, avec les 236 milliards supplémentaires, je parle de supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on est loin de la CNR vraiment de nombreux leviers existent afin de permettre à la sécurité sociale, d'être à l'équilibre, sans les Budgets qui pèsent sur l'hôpital, en particulier la logique redistributive et le principe de solidarité collective sont au coeur de l'histoire et du fonctionnement de la sécurité sociale, ils doivent être rappelés, ils doivent être renforcés. Oui, cet amendement propose une cotisation spécifique supplémentaire pour soutenir la dette sociale, en réalité, l'amendement telle qu'il est rédigé ne paraît pas opérationnelle en réalité, il n'est pas nécessaire à ce stade, les projections de la cadette permettant de respecter l'échéance de 2000 33 pour les stations l'extinction de la dette sociale, nous l'avons vu ensemble lorsque nous avons regardé précisément comment les déficits cumulés les robes et le FSV continue d'accumuler les déficits après 2024 donc on sera certainement obligé à un moment ou un autre, de se poser la question de de l'extinction de la dette ce sera un choix qui risque d'être affaire par les pouvoirs publics, en tout cas, par le gouvernement entre une nouvelle prolongation de la cadette ou l'augmentation des ressources qui lui sont affectés, mais en tout cas ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il faut en tout cas avoir cette préoccupation mais. Merci, monsieur le Ministre, ma ma vie. Défavorable je mais on voit le 742 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 12 qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté après cet article, l'amendement 777 Manama pour ce prix. Merci monsieur le président, il s'agit ici d'un amendement de repli qui va vous faire à tout ce plaisir puisqu'il perd, propose de mettre à contribution les actionnaires, notre groupe est le seul à s'être opposé à la création de la branche, perte d'autonomie qui repose uniquement sur les recettes fiscales et qui remet en cause excusez-moi de la sécurité sociale et le principe de la cotisation sociale, comme l'a dit tout à l'heure, ma collègue Laurence Cohen, nous proposons d'instaurer une contribution à 2 % sur les dividendes versés aux actionnaires, nous vous avons proposé de mettre à contribution les pas de privé lucratif, vous avez refusé, nous avons proposé de renforcer la fiscalité des actions gratuites, vous avez refusé, nous avons proposé d'augmenter la CSG, sur le capital, vous avez refusé, nous avons proposé de rétablir les cotisations patronales du CICE pour un montant de 25 milliards d'euros, vous avez refusé, nous avons proposé de supprimer les réductions Fillon de 26 milliards vous avez refusé, nous avons proposé de soumettre à cotisation sociale : les revenus financiers des sociétés. Vous avez encore refusé, nous avons donc a bon espoir que cette fois-ci, vous acceptez notre amendement dans tous les cas, vous ne pourrez pas nous reprocher de mettre en difficulté le financement de la Sécurité sociale ou que nous n'avons pas les moyens de recruter dans les EPHAD 300000 personnels, par exemple, puisque nous avons proposé près de 80 milliards d'euros de recettes supplémentaires que vous refusez. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Hé bien, ça va être assez simple en fait, nous refusons. Un avis défavorable, monsieur le Ministre, même avis. Donc je mais aux voix l'amendement 777 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté à l'article 13 le 811 1 Cohen. le gouvernement prévoit à l'article 13 de transférer 17,7 milliards d'euros à la 4S car il a fait le choix de financer les dépenses liées à la Covid 19 par la sécurité sociale au lieu de prendre en charge la dette par le budget de l'État, la loi du 7 juin 2020, qui a prolongé la durée de vie de la cadette afin qu'elle rembourse l'intégralité de la dette issue de la crise sanitaire a entériné une fuite en avant en fixant un objectif d'amortissement extrêmement court, au nom de la crédibilité sur les marchés financiers, la cadette, vous le savez, dispose de 3 sources de financement, la CRDS, une fraction de la CSG et l'abondement du fonds de réserve pour les retraites, ce qui représente un total compris entre 15 et 16 milliards d'euros, le gouvernement a donc fait le choix purement politique de se priver de quinze de 14 à 15 milliards issus de la CRDS et de la CSG, qui constituait la principale ressource disponible, sans augmentation des. Prélèvements obligatoires pour financer de réformes essentielles le Ségur de la santé, plus largement, l'hôpital public, si la dette sociale s'était éteinte, c'est parce qu'on avait serré la ceinture, si je puis m'exprimer ainsi, de l'hôpital public pendant plusieurs années on peut rouvrir le débat et faire marche arrière, mais nous refusons, vous l'avez compris depuis le début de ce débat, d'amputer le budget de la Sécurité sociale, j'ai moins d'humour que ma collègue mais je vous appelle à voter pour cet amendement. Merci madame la rapporteure. l'article 13, je le rappelle l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la caisse et de 17 7 milliards d'euros pour 2023 en fin 2023 la dette nette restant à amortir devrait s'élever à 104 54 virgule ce qui veut dire que 241,6 milliards d'euros ont été déjà amortie par la Cades S le transfert de la dette sociale prévue par l'article 1 de la loi du 7 août 2020 s'est poursuivie en 2022, à hauteur de 40 milliards d'euros venant réduire le besoin de financement induit par la crise sanitaire, je voulais rappeler ça parce que c'est important pour vous dire que l'article doit cet article doit obligatoirement figurer en fait dans la loi de financement de la Sécurité sociale, de prévision et d'information du Parlement et non un caractère normatif, c'est un article obligatoire, conformément aux dispositions de la loi organique que nous avions voté ensemble, de plus il était normatif amendement un fort risque d'inconstitutionnalité pour incompatibilité avec le respect de l'échéance organique du 31 12 2000 33 pour l'extinction de la dette sociale, c'est donc un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre, Même avis, donc je le mets aux voix le 811 avec 2 avis défavorables pieds. Pour qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2053 me madame Lubin. Nous proposons de supprimer le transfert de 17 milliards 700 millions d'euros de dettes à la Cades, le gouvernement a décidé de faire porter le coup de la Covid 19 à la sécurité sociale, une fois les dépenses effectuées par l'assurance maladie, notamment une partie de la dette Covid a été transféré à la cadette venant gonfler le montant de la dette que cette caisse est censé rembourser pourtant les dépenses liées au Covid ne relève pas intégralement des missions jardinières de la branche maladie, sa prise en charge par la dette de l'État nous paraît plus pertinente, si on prend en compte ces 17 milliards 700 millions d'euros, les administrations de Sécurité sociale dégage un fort excédent 0 5 point de PIB en 2022 0 8, en 2023, ça permettrait de mettre la sécurité sociale, ça permettrait à la sécurité sociale, d'être un accident et d'accroître les investissements dans le système de santé je crois me souvenir aller qu'à l'époque où ça a été fait, pas grand monde sur ces bornes étaient quand même d'accord avec ce transfert. Défavorable. Merci monsieur mise défavorable aussi. Je mets au voilà le 1053 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je Metz aux voix, l'article 13 qui. Pour qui est contre. Qui s'abstient-il était adopté après cet article trois amendements additionnel l'amendement 763 madame hommes. La loi 2019 828 du 6 août 2019, 2 transformations de la fonction publique, a assuré en son article 72, une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique depuis le 1er janvier 2020, selon le rapport annuel 2021 de la direction générale de l'administration de la fonction publique en 2020, seulement 428 ruptures conventionnelles ont été conclus dans la fonction publique toutefois dans le ministère de l'Éducation nationale sur les 1219 demandes de rupture conventionnelle déposées entre janvier et novembre 2020, seuls 296 ont abouti à une signature environ 24 % des démarches d'après habile bilan réalisé par le ministère, la part de refus est plus élevé que la part d'acceptation dans la fonction publique, la rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l'agent qui souhaite en bénéficier alors que l'on constate une recrudescence des démissions, des profs formés cet été pour la rentrée 2022 2023 les ruptures conventionnelles utilisées dans le secteur privé ne sont pas adaptés au fonctionnement des services publics, mais surtout, ces ruptures conventionnelles qui ne soient assujetties aux indemnités de rupture aux cotisations et contributions sociales aggrave le déficit de la Sécurité sociale, l'État refusant de compenser ces exemples sur de cotisations sociales, c'est la double peine pour la sécurité sociale qui se voit privés de recettes et de compensation financière par l'État pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons revenir sur cette disposition merci. Merci madame la rapporteure. Oui, chers collègues, c'est la double peine pour la sécurité sociale mais ce serait la double peine, surtout pour l'employé, qui perd son travail et donc cette indemnité qui est versée à la personne donc qui qui qui perd son emploi serait assez difficile à accepter, en période de fragilité, on peut le comprendre, donc c'est un avis défavorable. Si Monsieur le Ministre : avis défavorable aussi. Je mais aux voix l'amendement 763 et 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté de 764 un Oui, merci, monsieur le Président, j'ai déjà abordé la question et d'autres collègues l'ont fait de la du principe d'égalité salariale, vous savez que il était inscrit dans la loi depuis 1972 et que 50 ans plus tard, on en est toujours loin aujourd'hui, en 2022, les femmes gagnent en moyenne 15 8 pour 100 de moins que les hommes en France, selon les statistiques d'Eurostar, pardon, nous vous proposons donc que les entreprises de plus de 20 salariés dont le nombre de de salariés effectuant un temps partiel de moins de 24 heures égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l'entreprise soit soumise à une majoration de 10 % de leurs cotisations sociales, je pense que vous le savez, ce sont en majorité des femmes qui subissent les temps les temps partiels et donc, l'objectif est de limiter ce recours au temps partiel, quand il n'est pas choisie bien évidemment et quand il est subi, mais c'est en majorité un temps partiel subi, alors c'est vrai que régulièrement nous proposons cet amendement et qu'il est régulièrement refusé nous sommes opiniâtre, vous aussi, mais franchement, le Sénat devrait un peu bouger sur sa conception de l'égalité entre les femmes et les hommes, il existe des moyens aujourd'hui pour sanctionner les comportements les moins vertueux notamment la pénalité qui est prévu à l'article L. 22 42 tiré 8 du code du travail, laquelle peut aller jusqu'à 1 % de la masse salariale en cas de non-conclusion d'un accord ou d'un plan relatif à l'égalité professionnelle pour autant

donc il faut absolument y remédier, c'est tout le sens de notre amendement, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Oui, chers collègues, le le temps partiel, vous l'avez souvent dit correspond à des situations très différentes les unes des autres, en fait, il y a du temps partiel subi, et il y a aussi du temps partiel choisi et puis il y a aussi des secteurs d'activités qui peut pas faire autrement que de multiplier finalement les propositions de temps partiel, donc en réalité, tout ça pour vous dire que c'est un avis défavorable, parce que une telle sanction qui est indistincte de ces cas différents, en fait, ne paraît pas. Merci, Monsieur le Ministre, même avis même avis défavorable Madame Cohen. Moi, je suis désolé, hein, l'heure est tardive, ou c'est tôt le matin mais je trouve que le débat mérite d'être poussé

stupéfaite par les arguments qui nous sont opposés Kant, on essaye de, de, de parvenir à l'égalité salariale, je suis toujours stupéfaite parce que sont toujours alors oui mais peut-être il y a des temps subie mais ils ne sont pas si Subic que ça mais enfin, on est sur le budget de la Sécurité sociale je crois, mes chers collègues, ou alors je me trompe mais on a tous dans nos départements des iPads on a tous dans d'autres départements, des aides à domicile qui viennent à nos permanences, je ne crois pas être la seule à avoir cette fréquentation à mes permanences et qui se plaignent, je pense notamment aux aides à domicile de du temps fractionner les courses qu'elle doive faire pour arriver à, à aller voir telle ou telle patients et si j'élargis, pas seulement au monde de la santé mais mais je on peut parler aussi des caissières et cetera, c'est la même chose. Et vous ne faites rien. Vous n'accepter aucun de nos amendements et vous n'en proposer aucun. Et en fait tout va bien dans le meilleur des mondes, alors je sais bien que dans le Sénat, on n'a pas encore la parité qu'on en est bien loin, qu'il faut vraiment à chaque fois. à faire beaucoup d'efforts pour essayer de gagner un nombre de femmes opposition électives quand on est, on n'a pas des listes, mais quand même, vous pourriez être un peu intéressé à l'égalité à l'émancipation de notre société et donc ça serait une preuve d'ouverture du Sénat qui manque que quelle que soit l'heure à laquelle nous posons ces arguments, donc je vous appelle à méditer, à cette heure tardive, et peut-être à changer votre position.

Merci monsieur le président, notre groupe dépose chaque année cet amendement qui est vécu comme une injustice pour les hôpitaux et les et les pas de public actuellement la majorité des établissements publics bénéficient d'une exonération de la taxe sur les salaires, ainsi les collectivités territoriales, les universités, les centres d'action sociale, les régies publiques l'Établissement français du sang et Jean ça, j'en passe sont exonérés de cette taxe, nous demandons par cohérence que les hôpitaux soient exonérés de la taxe sur les salaires, tout comme les épate qui contrairement aux pas de privé ne bénéficient pas des exonérations du CIT s la suppression de cette taxe permettrait de redonner plus de 5 milliards d'euros aux hôpitaux qui en ont besoin en 2019, la ministre de la Santé avait rejeté notre amendement car les services du ministère, travailler sur une refonte du barème en 2020, celle-ci avait rejeté notre amendement car un rapport sur le sujet était en cours de rédaction en 2021, celles-ci avait rejeté notre amendement car les recettes de la taxe sur les salaires étaient réinjectés dans les différentes branches de la Sécurité sociale et que notre amendement entraînerait une réduction des crédits des autres branches de la Sécurité sociale, nous avons hâte de connaître la vie en 2022 du nouveau ministre de la Santé, mais d'ores et déjà, il est évident que si le gouvernement rétablissez les cotisations sociales et stopper les exonérations de cotisations on arrêterait la fiscalisation de la Sécurité sociale et les allers-retours budgétaire dont la Cour des comptes elle-même dénoncé la klongs complexité illisible de la fiscalité du financement de la Sécurité sociale, en attendant ce sont 5 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux, quand les personnels sont au bord de l'épuisement ce serait un signe positif alors en droit d'adopter cet amendement, je vous remercie. Eh bien, malheureusement, la réalité c'est que nous n'avons pas changé hein depuis l'année dernière et et que c'est la même punition en quelque sorte puisque c'est un avis défavorable en fait, les hôpitaux et les Ephad public ne sont pas des collectivités, vous l'avez souligné et donc ils ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, en outre, une telle mesure représentait représenterait une perte conséquente pour la sécurité sociale, alors vous parlez des de toutes les branches, mais c'est surtout en particulier, la branche vieillesse qui serait en tout cas pénalisé donc qui devrait en plus subir de forts déficits, les années à venir, c'est pas le moment de leur enlever cette branche à cette branche vieillesse cette taxe sur les salaires. Même avis pour Monsieur le Ministre. Donc je mais aux voix l'amendement 767 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 14 qui est, pour qui elle compte qui s'abstient, il est adopté, article 15 Madame Cohen a demandé la parole. On s'arrête pas Madame Cohen. je croyais qu'ont continué jusqu'à une heure. je remercie la rapporteure. Général pour nous répondre toujours avec précision même sur six je suis en désaccord avec ce qu'elle nous dit alors, avant d'entamer les amendements sur l'article 15 concernant l'approbation du rapport sur l'évolution pluri-. Du financement de la Sécurité sociale, je voudrais faire le lien avec l'examen la semaine dernière de la loi de programmation des finances publiques, je pense notamment à son article 17 qui fixe le calendrier, le cadre financier des administrations, de la sécurité sociale pour les années 2023 2027, le gouvernement prévoit ainsi que les dépenses des hôpitaux progresseront de 4 1 pour 100 en 2023, de 9 % en 2024 et de 8 % en 2025, soit une hausse des dépenses de santé inférieurs. Ah l'évolution naturelle des dépenses estimées par la commission des comptes de la Sécurité sociale, qui je vous le rappelle, est de quatre. Pour % est inférieur aux prévisions d'inflation, autrement dit, non seulement le gouvernement ne prévoit pas d'augmenter le budget des hôpitaux pour cette année mais il ne prévoit pas d'augmenter le budget d'ici 2025, tout au contraire, il va Real il va réaliser des économies sur le dos de la santé, alors quand on sait. Quel est l'état de notre système de santé publique, on ne peut que s'opposer à cette politique, mais malheureusement, ici au niveau du sénat, hé bien il y a une connivence entre la politique du gouvernement et celle de la droite, et c'est ce qui fait que la politique passe et que les les hôpitaux continuent à être à bout de souffle, les personnels exténué et qu'effectivement nous au niveau du groupe communiste républicain et citoyen, on continue à porter leur parole, même quand il est une heure du matin. Oui merci monsieur le président, alors, enfin, Madame Cohen, nous allons pouvoir nous rejoindre sur le dernier amendement qui est en fait communs cas c'est la suppression de l'article 15. Et c'est effectivement une une comment approbation de la proposition de l'annexe.

on revient à ce qu'a dit aussi, le Haut Conseil des finances publiques en fait il y a des effets importants supposée des réformes comme l'assurance chômage, l'apprentissage, les retraites qui ne sont pas en fin de compte, pris en compte, sinon dans un un peu dans l'annexe mais on connaît pas les modalités, on ne connaît pas les impacts on connaît pas le calendrier, on ne connaît pas, bref, les conditions dans lesquelles ces ces, ces, ces réformes seront mises en place, donc ça rend fragile la trajectoire des finances publiques, on trouve aussi qu'il y a une provision insuffisante concernant la prise en compte des dépenses Covid pour l'année, un milliard d'euros, c'est quand même insuffisant par rapport à ce qu'on a vu dernières années même si on sait que, on vit avec, désormais, l'inflation est élevé en 2003, donc ça fait une hausse des dépenses, là encore, il semblerait que ce ne soit pas assez pris en compte, je voudrais aussi rajouter que le Haut Conseil des finances publiques, a observé que les dépenses d'assurance-maladie dans le Champ de l'Ondam, se sont inscrites en progression sensiblement moins rapide que le PIB ce qui s'est rarement produit par le passé, alors pourquoi ça se produirait là une absence donc compléter délibérée de plan stratégique, c'est la 2ème raison hein qui nous amène à à supprimer cet article donc la dimension pluriannuelle doit donner une visibilité, alors non seulement comptable mais aussi, et stratégique au Parlement, et au-delà à l'ensemble des acteurs de la sécurité sociale et j'ai envie de dire à la société toute entière et c'est pas ce qu'on veut. Trouve dans cette annexe B comme Madame Cohen et ses collègues, je propose de supprimer cet article 15. Merci de 1100 va madame pour ce prix. Hé bien, voilà la bonne parole de la fin non oui. Oui, on va se retrouver l'annexe B prévoit la trajectoire de recettes et de dépenses de la Sécurité sociale dans les prochaines années son alinéa 25, souligne que le déficit de la branche vieillesse et du FSS sera directement. ouais, ouais, ouais, je crois, on est fatigué. Pourtant, on dit qu'on n'est pas fatigué, hein non allez cet article 15 propose madame évidemment d'approuver le rapport sur l'évolution pluri-annuel du financement de la Sécurité sociale, constituant l'annexe B du Plfss pour 2023 la trajectoire présenté par l'annexe B

ce ralentissement de l'Ondam va entraîner une augmentation d'objectif de seulement de 6 7 milliards d'euros. Par an alors que les besoins sont estimés à 10 milliards d'euros supplémentaires pour tenir compte simplement de l'évolution naturelle des dépenses de santé, ce chiffre ne tient pas compte de la nécessité du rattrapage du retard accumulé en matière d'investissement de recrutement et de fonctionnement concernant la sincérité des prévisions de cette évolution pluriannuelle je rappellerai également que le Haut Conseil des finances publiques

par rapport aux besoins des hôpitaux, nous refusons la poursuite des politiques d'austérité en matière de santé pour c'est des raisons nous demandons la suppression de l'article, comme vous l'avez fait avec votre amendement numéro 45 madame la rapporteure générale. Merci monsieur le le président même la la rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, avis défavorable à la à la à la suppression de l'annexe B pour 3 raisons: la première, c'est que le Haut conseil aux finances publiques, il a jugé que les les prévisions du gouvernement en matière de masse salariale et d'inflation était crédible et s'il a soulevé un problème d'incertitude et d'aléas, il est lié à la conjoncture, mais pas au à des problématiques liées à la prévision et au chiffre retenu par le gouvernement. Mais il vous appartient évidemment de de contester ces ces prévisions et ce qui m'amène à mon 2ème point peut-être auriez-vous

alors le texte n'est pas conforme à la Constitution et donc sans doute utile fallu amender cette annexe B pour qu'ils correspondent aux prévisions que que vous jugez pertinente mais mesdames et messieurs les les sénateurs, la 3ème, raison pour laquelle je voudrais vous demander de retirer cet amendement c'est que sachant que mercredi dernier, vous avez voté cette trajectoire de la sécurité sociale en votant la loi de financement. Hé ouais. Certes, en présence de mon éminent collègue Gabriel Attal alors vous me verriez bien peiné si ce soir en ma présence vous rejette cette trajectoire de la Sécu. Voilà. Merci, monsieur le Ministre, donc je mais ou vois ces deux amendements identiques. Alors moi c'est mouillé. Oui, très rapidement Monsieur présent du tardive, juste une remarque par rapport à l'intervention de Monsieur le Ministre, vous avez certainement suivi les débats et l'argumentaire qui a fait qu'on a pu voter la semaine dernière, donc le les, les, les résultats financiers, on a eu un argumentaire basé principalement sur le doute sur la non-sincérité sur la capacité d'avoir des chiffres réels sur la capacité d'avoir une vision et donc, par cohérence, nous avons voté ces textes-là et donc aujourd'hui on vient à traduire ce doute, cette capacité à avoir cette vision et donc quelque part, je pense que ce vote est formel : il est nécessaire et c'est peut-être un signe que vous devrez faire remonter auprès du gouvernement.

Et nous passons un article additionnel après l'article 15 le l'amendement 1054 madame Dubin. Oui, c'était un amendement qui prévoit que tout nouveau dispositif d'exonérations sociales est accompagnée de la suppression d'un dispositif existant, pour un montant équivalent, nous partons d'un constat simple : au cours des 1er et 2ème trimestres 2021, le taux de marge des entreprises s'est envolé, aux alentours de 36 % selon l'Insee, son plus haut niveau depuis 1949 date à laquelle l'institut a commencé la mesure de ce ratio en même temps, le montant total des aides publiques reçues par les entreprises atteint 8 4 % du PIB, selon le chercheur de l'IRES si l'un des plus haut taux de l'OCDE, notre proposition est donc simple : arrêter d'embêter les finances publiques avec des dispositifs d'exonération peu efficace écoute. Merci madame la rapporteure. rentrer ce soir, mais en réalité, la dernière fois, nous avons voté un repère, une référence, or là, c'est un acte politique et nous refusons cette enfin cette trajectoire qui nous semblent manquer en fait de réalités de réalisme et surtout d'un manque de stratégie. Pour répondre à ma collègue, je dirais que c'est un avis défavorable, parce qu'une telle pétition de principe sans effet normatif aurait mieux trouver sa place au sein de la loi de programmation des finances publiques, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, chers collègues, et je pense que ça aurait toute sa place, donc c'est un avis défavorable. Merci mais même avis pour Monsieur le Ministre. Donc je mais on voit le 1054 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix la 3ème partie du projet de loi, je rappelle que l'application de l'article 47 bis ah du règlement lorsque le Sénat de te pas les dispositions de cette partie, la 4ème partie de ce projet de loi est considéré comme rejeté, y a-t-il des demandes d'explications de vote. Je n'en vois pas donc je mais aux voit la 3ème partie du projet de loi il y a un scrutin public. Donc, le scrutin est ouvert.

Tout est clos. Ah du scrutin 36 Nombre de votants : 343 Nombre de suffrages exprimés 343 pour l'adoption 252 contre 91, le Sénat a adopté. Madame de roche la présidente. Oui, pour remercier les collègues pour ces 2 jours de débats remercier qu'on ait puis qu'on ait pu grâce à votre présence à une forme de discipline, même s'il y a eu beaucoup de beaucoup d'interventions, nous permettent de terminer sa 3ème partir, merci Monsieur le Ministre, pour la qualité de ses réponses et et vraiment remercier également bien évidemment la séance, les administrateurs et nous vous disons à demain après-midi. Mais rapporteur. Oui, si vous me le permettez, monsieur le président, puisque mon travail va s'arrêter là, en tout cas auprès de madame la présidente de la commission des affaires sociales, remercier l'ensemble des ministres qui sont venus pendant ces 2 jours, remerciez évidemment l'ensemble de la commission qui a été assez indulgente, on a eu le texte quand même très, très tard, il a fallu travailler très, très tard, et c'est vrai que je je comprends parfois la frustration de mes collègues quand on on abat l'ensemble des des amendements de façon aussi rapide, en tout cas je pense qu'on a déjà eu un débat, on a rétabli la partie hein et de qui était quand même escamoté, qui a été escamotée à l'Assemblée nationale, je voudrais remercier en particulier David Bonnet qui travaille à mes côtés, il y a aussi comment Douglas petit et puis les autres administrateurs qui ont été sur certains amendements, aussi très actif, merci à Delphine d'emmener toute cette équipe merveilleusement bien, en tout cas merci à tous et puis on va continuer de travailler pendant les jours prochains, donc. à demain, merci. Merci, mes chers collègues, je vais lever la séance, nous avons examiné 134 amendements au cours de la journée, il en reste 426 à examiner sur ce texte prochaine séance mercredi 9 novembre à 15 heures les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.